vise à diviser par deux les crédits de l'expérimentation des emplois francs et à les porter à 90 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 5,8 millions d'euros en crédits de paiement. Trois raisons justifient son dépôt. La première est le coût excessif de l'expérimentation proposée par le Gouvernement, quasiment un demi-milliard d'euros en autorisations d'engagement, pour une expérimentation d'un an et demi. À titre de comparaison, l'expérimentation « Zéro chômage de longue durée », d'une durée de cinq ans, coûtera seulement 18 millions d'euros en 2018. La deuxième raison concerne les doutes sérieux sur l'efficacité des emplois francs. Le Gouvernement, échaudé par l'échec de l'expérimentation en 2013 et 2014, qui avait vu moins de 300 contrats de signés, a refusé de prévoir des critères d'âge et de diplôme pour verser l'aide. Il n'a pas ciblé non plus de secteurs d'activité prioritaires. En agissant ainsi, le risque est grand de faire apparaître des effets d'aubaine. Or je vous rappelle que c'est justement ce risque qui a justifié la suppression, par le Gouvernement, des emplois aidés dans le secteur marchand. La troisième raison est l'absence d'information sur des paramètres décisifs de l'expérimentation, comme le nombre prévisionnel d'embauches en CDI et en CDD. L'impression se dégage d'un dispositif conçu tardivement, dans la précipitation, une « danseuse » en quelque sorte, qui ne permet pas au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause. Au final, cet amendement ne tend pas à supprimer l'expérimentation. Bien au contraire, il vise à l'encadrer et à mettre le Gouvernement face à ses responsabilités, en agissant par voie réglementaire s'il le souhaite.

de la mission « Travail et emploi », d'accélérer la mise en oeuvre des emplois francs, qui constituent un engagement important du Président de la République en faveur des quartiers populaires. Aussi un dispositif d'expérimentation sera-t-il déployé dès 2018 sur plusieurs territoires. Pour rappel, le dispositif permettra à une entreprise ou à une association, où qu'elle où qu'elle soit située sur le territoire national, de bénéficier d'une prime pour l'embauche d'une personne résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville, à hauteur de 5 000 euros par an pendant trois ans maximum en contrat à durée indéterminée et à hauteur de 2 500 euros par an durant deux ans maximum pour un contrat à durée déterminée de plus de six mois. Le Président de la République a annoncé, le 15 novembre dernier, la liste des territoires retenus pour l'expérimentation. Le choix a été fait de retenir des territoires emblématiques et représentatifs de la diversité des quartiers prioritaires de la politique de la ville : la Seine-Saint-Denis, l'agglomération d'Angers, l'agglomération Val de France et celle de Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise, le territoire Grand Paris Sud englobant Grigny et Évry, une partie des métropoles de Lille et de Marseille. Ces territoires représentent environ 25 % des demandeurs d'emploi en quartier prioritaire de la politique de la ville. Le choix a donc été fait d'assurer une expérimentation de grande ampleur et en même temps concentrée sur quelques territoires, le tout afin d'assurer une réelle appropriation du dispositif par les acteurs locaux. Ce choix ainsi que l'élargissement des critères d'éligibilité et le relèvement du montant de l'aide pour le rendre plus incitatif permettront à la mesure, dès sa phase d'expérimentation, d'avoir un effet réel sur les discriminations territoriales. La mesure est La mesure est conçue dans un objectif d'insertion durable dans l'emploi de droit commun. Il ne s'agit pas ici de créer des passerelles hypothétiques vers l'emploi, mais d'assumer une politique d'emploi insérée de manière naturelle dans les parcours professionnels et le tissu économique existant. Enfin, le choix de passer par une première étape d'expérimentation permettra de conforter et, le cas échéant, d'adapter les conditions d'efficacité du dispositif, en vue de sa généralisation à l'horizon de 2020, comme le prévoit la trajectoire pluriannuelle des crédits de la mission « Travail et emploi ». La remise au Parlement d'un rapport d'évaluation est prévue au plus tard le 15 septembre 2019.

est ainsi libellé : La parole est à M. Yves Daudigny. Les structures d'insertion par l'activité économique permettent aujourd'hui à 140 000 personnes chaque mois d'être employées, accompagnées et formées en vue de leur retour sur le marché du travail de droit commun. Elles sont, pour ces personnes éloignées de l'emploi et souvent disqualifiées aux yeux des employeurs par la durée de leur chômage et les problématiques sociales qu'elles peuvent rencontrer, l'un des seuls moyens d'accéder à court terme à l'emploi et d'enrayer la spirale de l'exclusion. Les personnes durablement éloignées du marché du travail sont aujourd'hui au nombre de 2,5 millions. Pour empêcher que cet éloignement soit définitif, pour empêcher que d'autres personnes actuellement privées d'emploi basculent dans cette situation, il nous paraît essentiel d'augmenter leurs possibilités d'emploi, l'augmentation du nombre de postes d'insertion au sein des structures de l'insertion par l'activité économique. Le présent amendement a donc pour objet de doter l'action n° 02 Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail du programme 102 Accès et retour à l'emploi » de 60 millions d'euros supplémentaires, destinés au financement de postes d'insertion par l'activité économique. Il vise, en conséquence, à diminuer

Ces structures jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement vers l'emploi des personnes très éloignées du marché du travail. C'est pourquoi le projet de loi de finances pour 2018 prévoit déjà une augmentation des crédits consacrés à l'IAE de l'ordre de 30 millions d'euros,

lequel reste limité notamment pour ce qui concerne les ateliers et chantiers d'insertion, les ACI, en raison de la complexité de l'articulation entre les financeurs. Il s'agira de rendre plus fluide l'accès aux différentes formations. Le plan d'investissement des compétences, le PIC, constituera à cet égard un levier important. L'avis est donc défavorable.

qui travaillent dans ces structures. C'est pourquoi cet amendement vise à abonder de 50 millions d'euros les crédits de l'action n° 01, Amélioration du service public de l'emploi, du programme 102 « Accès et retour à l'emploi », en diminuant d'autant les crédits de l'action n° 04,

outre, cette réduction est compensée par la dynamique de la contribution de l'UNEDIC. Assise sur la masse salariale, cette augmentation est évaluée à 70 millions d'euros en 2017 et 2018. La baisse de la subvention de Pôle emploi se justifie par l'effort transversal demandé aux opérateurs publics. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

offrent des solutions dynamiques de création d'emplois. Il faut désormais mettre en oeuvre le contrat de développement responsable et performant du secteur adapté, signé en mars 2017. Cet amendement vise à augmenter le budget dédié à la subvention spécifique qui vient en complément des aides au poste pour les entreprises adaptées, qui emploient à 80 % des personnes en situation de handicap. La subvention spécifique est destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée. Elle n'avait pas été augmentée au cours de la précédente législature. La baisse de 22 % prévue pour 2018 est préjudiciable. Cet amendement est directement lié à la mesure prévoyant la baisse de 7,59 millions d'euros de la subvention spécifique et la création de 1 000 aides au poste supplémentaires pour l'année 2018. la personne en situation de handicap en recherche d'emploi possède un faible niveau de qualification et que sa durée moyenne d'inactivité est supérieure de 200 jours à celle du public valide. La création de 1 000 aides au poste ainsi que la baisse de 7,59 millions d'euros de la subvention spécifique induisent, en conséquence, une augmentation du budget dédié à la subvention spécifique de 9,37 millions d'euros. Il est proposé de financer cette augmentation par des transferts de crédits.

trouve un emploi dans une entreprise adaptée, cela représente une économie moyenne de 10 000 euros pour la collectivité.

d'emploi des personnes en situation de handicap. Comme le précédent, le présent amendement vise à compenser les baisses de crédits envisagées pour l'aide spécifique et à prendre en compte, dans le même temps, la création de 1 000 aides

Ces 8 millions d'euros sont prélevés sur l'action n° 16 du programme 155. Le renforcement du soutien financier à l'aide au poste permettra logiquement qu'une économie de même montant soit réalisée sur les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail.

pris lors du Comité interministériel du handicap visant à changer le regard sur le handicap et à construire une société plus inclusive. Cet amendement est directement lié, d'une part, à la baisse de 8 millions d'euros du montant

original d'entreprises ordinaires inclusives. À la suite de ce débat, Mme la ministre du travail a demandé à son cabinet d'échanger et de se concerter avec l'ensemble des représentants du secteur, notamment pour s'assurer de leur engagement à travailler dès le début de 2018 sur des modalités rénovées et simplifiées de financement et de pilotage des entreprises adaptées.

trouver les voies, par l'innovation notamment, du développement de l'emploi durable des personnes handicapées dans les entreprises adaptées comme dans les autres entreprises et accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre de ces nouvelles orientations. À ces conditions et au vu des travaux de concertation à conduire, nous sommes prêts à reporter la mise en oeuvre

personnes handicapées. Cet effort, supérieur à celui consenti lors des derniers exercices, se traduira par une augmentation de 8 millions d'euros des crédits dédiés au financement de ces aides au poste. Celles-ci seront financées selon les règles actuelles, soit à hauteur de 80 % du SMIC, dans l'attente des inflexions envisagées pour 2019.

par les collectivités et de 15 % par le FSE. En accord avec les priorités fixées par le Gouvernement, il est proposé de rétablir les autorisations d'engagement et les crédits de paiement déployés sur l'année 2017, soit 21 millions d'euros. Il convient ainsi de diminuer les crédits de l'action 01, sous-action n° 02, Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés, du programme 103, « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », de 9 millions d'euros et de les transférer vers l'action n° 01, sous-action n°

Nous ne lâcherons pas prise, car la réponse qui nous a été apportée en octobre, puis aujourd'hui- réponse brève et cassante -, n'épuise absolument pas la question. On nous renvoie à Pôle emploi et aux missions locales, qui rempliraient le rôle de guichet unique initialement attribué aux maisons de l'emploi. Or cela fait dix ans que les maisons de l'emploi font autre chose elles ont un rôle d'ingénierie territoriale ; elles remplissent des missions de définition des besoins sur le bassin d'emploi qui est le leur ; elles animent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; elles travaillent en direct avec les entreprises ; elles soutiennent de jeunes créateurs d'entreprise ; elles animent aussi le réseau local de facilitateurs de la clause sociale d'insertion, et tant d'autres choses tout ce que vous louez en vue de mettre en place le plan d'investissement des compétences. Ce sont autant de missions que ne remplit pas Pôle emploi, et pour cause ! À la demande des élus locaux, des acteurs de terrain, et même de Pôle emploi, de l'emploi, souples et pragmatiques, sont devenues une plateforme collaborative, complémentaire à Pôle emploi. La ministre du travail a fait savoir qu'elle souhaitait travailler sur l'emploi avec les élus locaux. Faites-le ! Ce sont eux qui portent ces maisons. Elles existent par la volonté des élus locaux de participer, aux côtés de l'État, à cette belle idée lancée par Jean-Louis Borloo. Écoutez Alain Juppé, Martine Aubry, Johanna Rolland, Georges Képénékian, et tant d'autres élus locaux ! Ne laissez pas, une fois de plus, nos collectivités en rase campagne, comme dans le dossier des contrats aidés par exemple. Si vous persistez dans cette coupe claire, peu de maisons de l'emploi se relèveront, et les territoires les plus fragiles seront encore durement pénalisés. Je suis certaine que votre souhait n'est pas d'institutionnaliser la fracture territoriale dans vos politiques publiques.

aux orientations fortes du Gouvernement : analyse des besoins des entreprises, des compétences souhaitées, construction de plans de formation, gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences, ou GPTEC. également que le coeur de l'action des maisons de l'emploi s'est progressivement centré sur la GPTEC, levier tout à fait adéquat pour faire face aux nouveaux défis des territoires en termes de mutations économiques pour mieux valoriser les ressources territoriales, assurer leur correspondance avec les besoins, prévoir leur adaptation aux évolutions à venir. En outre, les maisons de l'emploi animent la mise en oeuvre de la clause sociale d'insertion sur le territoire, qui est sans doute un dispositif performant en matière de retour à l'emploi au niveau national, dispositif lancé en 1995 par les plans locaux pour l'insertion et l'emploi. Ce sont 433 facilitateurs de la clause qui animent sur l'ensemble du territoire français ce dispositif, financé à hauteur de 20 % par par l'État au titre des maisons de l'emploi et de 80 % par d'autres financeurs, dont 40 % par les collectivités. Affaiblir encore davantage les maisons de l'emploi en diminuant leur budget serait donc contre-productif pour les territoires et reviendrait à se priver de compétences qui sont disposées à contribuer à la réussite des enjeux nationaux. Notre amendement vise donc à diminuer les crédits de l'action n° 01, sous-action n° 02, du programme 103, de 9 millions d'euros et de les transférer vers l'action n° 01, sous-action n° 02, Coordination du service public de l'emploi, du programme 102, « Action et retour à l'emploi ». La parole

des élus locaux sensibles aux équilibres de nos territoires, je l'entends bien. Toujours est-il que, depuis 2009, force est de constater que les maisons de l'emploi n'ont plus la même utilité.

L'idée initiale visant à faire un guichet unique a été battue en brèche en 2008, avec la création de Pôle emploi. Aussi les missions financées par l'État se limitent-elles depuis 2013 aux deux axes suivants, qui n'intègrent pas l'accueil du public, souvent mis en avant

de 86 millions en 2010 à 21 millions d'euros en 2017. La réduction des crédits de l'État n'est donc pas une question nouvelle. Dans le prolongement de ces évolutions et au vu des besoins prioritaires portés par la mission « Travail et emploi », le choix a été fait de poursuivre jusqu'à son terme le retrait du financement du fonctionnement de ces structures par l'État. Un effort a toutefois été consenti en première lecture par l'Assemblée nationale, avec un abondement de 1,5 million d'euros du budget des maisons de l'emploi permettant de réduire la baisse du financement de l'État à 43 %, au lieu des 50 % prévus initialement lors de cette année de transition. Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, que la réduction de la part financée par l'État ne signifie pas nécessairement la fin des maisons de l'emploi, celles-ci pouvant bénéficier d'autres financeurs pour leurs actions. À ce titre, le Gouvernement précise également que des financements pourront être obtenus dans une logique de soutien non plus à un réseau,

Les maisons de l'emploi permettent d'améliorer la lisibilité des structures qui interviennent sur le territoire et facilitent leur mise en relation. Les nombreux partenariats avec les collectivités territoriales, les acteurs du développement économique, ceux de la formation et de l'insertion, les organisations professionnelles,

Les jeunes occupent de vrais emplois qui valorisent et permettent d'accroître leurs compétences. Dans le secteur non marchand, ils contribuent à apporter des services à la collectivité et donc à dynamiser les territoires en prenant en compte des besoins mal satisfaits,

madame la ministre le Gouvernement vous a d'ores et déjà transmis, le 8 février 2017, un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir. En outre, le ministère du travail réfléchit actuellement à une nouvelle évaluation du dispositif. Ces amendements étant sans objet, l'avis est donc défavorable.

de la recherche, des études et des statistiques, et un volet qualitatif, confié à une équipe multidisciplinaire intégrant notamment le Centre d'études de l'emploi et du travail, recruté pour appel à projets. Ce travail d'évaluation devrait se conclure d'ici à la fin de l'année. Au vu des travaux de ce comité, un rapport d'information sur l'évaluation du plan n'est pas opportun

ainsi proposé de limiter la dérive en la matière, en maintenant le nombre de contrats aidés sous le nombre de titulaires ou de contrats de droit commun.

À ce stade, il ne me paraît donc pas nécessaire d'inscrire ce point dans la loi : avis défavorable.

la mission « Culture », mais également les crédits de la recherche culturelle, ceux qui sont consacrés au livre et aux industries culturelles et, enfin, la part des concours financiers aux collectivités locales destinés aux bibliothèques. La mission « Culture », plus spécifiquement, est en augmentation de 40 millions d'euros en crédits de paiement. Elle regroupe les crédits de la politique culturelle consacrée aux patrimoines, à la création artistique, à l'enseignement supérieur de la culture et à l'accès à la culture. Elle comprend également les fonctions de soutien du ministère

15,4 millions d'euros sont reventilés vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », mais l'éducation artistique et culturelle bénéficie également de 35 millions d'euros de mesures nouvelles, en crédits de paiement. Cette priorité s'accompagne d'objectifs ambitieux en matière d'accès des jeunes publics à la culture, de réalisation d'un parcours complet d'éducation artistique et culturelle dans ses trois composantes- la pratique artistique, la fréquentation des oeuvres et la rencontre avec les artistes -et, enfin, d'acquisition de connaissances dans le domaine des arts et de la culture. Le développement des pratiques artistiques et culturelles implique une collaboration renforcée entre le ministère de la culture et celui de l'éducation nationale. Les crédits de la mission contribueront, par exemple, à l'amplification du plan du ministère de l'éducation nationale en faveur des chorales. Les crédits supplémentaires dédiés en 2018 à l'éducation artistique et culturelle permettront également d'approfondir des dispositifs existants, tels que les contrats territoire lecture. Les établissements publics opérateurs de la mission contribuent, eux aussi, à des actions d'éducation artistique et culturelle, pour un montant évalué au total à 30 millions d'euros. Le rôle de ces opérateurs est essentiel ; ils mènent, à leur niveau, des actions souvent très efficaces en la matière. C'est le cas par exemple de la Philharmonie de Paris,

veux souligner un second point positif pour la mission « Culture », en 2018 : l'effort budgétaire est maintenu, voire renforcé, pour le soutien à l'entretien et à la restauration des monuments historiques. Un effort particulier est fait à destination des collectivités locales à faibles ressources financières ; une grande partie des 43 000 monuments historiques est en effet localisée sur le territoire des communes de moins de 2 000 habitants. Par ailleurs, on constate un désengagement progressif des départements du financement des opérations de restauration ; un fonds de 15 millions d'euros, réparti entre les DRAC et géré par elles, permettra une participation financière de l'État là où les régions décideront de financer des projets. Ce fonds s'inscrit dans le cadre de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, que vous avez présentée le 17 novembre dernier. Celle-ci comprend également la mission confiée par le Président de la République à Stéphane Bern, qui consiste à identifier le patrimoine immobilier en péril et à chercher des solutions innovantes pour assurer le financement des travaux indispensables. Cette mission n'implique pas de coût budgétaire dédié, mais les services du ministère de la culture chargés des monuments historiques seront mobilisés. Une plateforme électronique a été mise en ligne sur le site du ministère de la culture pour que les monuments concernés soient déclarés. L'analyse et la cartographie du patrimoine en péril seront réalisées avec le concours de ces services. Par nous avons à nouveau mis en évidence cette année la nécessité d'une vigilance particulière sur les nombreux chantiers immobiliers d'envergure du ministère et de ses opérateurs. Ces projets concernent l'ensemble des programmes de la mission- le Grand Palais, la Cité du théâtre, la relocalisation du Centre national des arts plastiques à Pantin -ou encore les nombreux schémas directeurs, tels que celui de l'établissement public de Versailles ou celui du château de Fontainebleau. Pour chacun de ces chantiers, il est nécessaire de suivre avec attention le respect des coûts et des délais. Je conclus en disant que, en 2018, l'effort budgétaire pour la culture est maintenu. Le soutien au patrimoine et à la création n'est pas remis en cause par la priorité donnée à l'accès à la culture pour tous, ce dont nous pouvons nous satisfaire. je vous indique, pour finir, que la commission des finances a suivi la proposition de vos rapporteurs spéciaux et vous propose d'adopter les crédits de la mission, sans modification. La parole est à M. le rapporteur spécial. Monsieur

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la priorité de ce budget est claire : la démocratisation culturelle, l'accès de tous les publics à la culture ou encore l'éducation artistique, appelons cela comme l'on veut.

Ce pass doit être l'aboutissement du parcours d'éducation artistique et culturelle. La mise en oeuvre du pass culture sera à suivre avec attention ; le périmètre et les modalités de son financement doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie en 2018. Un montant de 5 millions d'euros de crédits de paiement est d'ores et déjà inscrit c'est beaucoup pour une préfiguration, mais cela permettra de financer les études et la conception d'un outil informatique innovant. Il faudra bien sûr s'inspirer de ce que font déjà certaines collectivités ou de l'expérience italienne. Le coût estimé est de 140 millions d'euros par an pour l'État, mais cela représente le tiers du coût total, puisque la participation des distributeurs ou des grands acteurs d'internet est envisagée par le Gouvernement. Avec l'ouverture des bibliothèques le dimanche, cette mesure met la question des publics au coeur de la politique culturelle. À ce titre, le choix d'un indicateur de performance centré sur les scolaires, et notamment sur le fait qu'ils bénéficient d'un parcours complet, est aussi un signal fort en lien avec l'éducation.

fonds propres, c'est-à-dire grâce au mécénat et, surtout, à la vente de l'actuel site du Conservatoire. L'objectif, pour les établissements concernés, est aussi de pouvoir absorber le coût de fonctionnement de ces nouveaux locaux par des recettes supplémentaires et par les économies de gestion réalisées. Toujours en matière de diffusion, nous avons mis en évidence, lors de la présentation de notre rapport spécial à la commission des finances, la nécessité de rester vigilant quant à la réponse apportée aux demandes des établissements culturels dans le cadre du Fonds d'urgence pour le spectacle

pour le ministère de la culture. Les crédits de la mission « Culture » sont donc préservés en 2018, le président Éblé vient de le rappeler. J'ajoute que la prévision triennale présentée dans la loi de programmation inscrit également cette mission dans une progression sur la période 2018-2020, avec une augmentation de 50 millions d'euros sur trois ans. C'est donc un effort qui n'est pas simplement fourni en 2018 mais qui sera prolongé.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, incontestablement, le patrimoine connaît, ces derniers mois, un net regain d'intérêt ; les membres de la commission et moi-même Les récents rapports de Martin Malvy et d'Yves Dauge n'y sont sans doute pas étrangers. Votre souhait, madame la ministre, de faire des politiques patrimoniales un levier tant de l'accès du plus grand nombre à la culture que de que de l'attractivité des territoires et de la revitalisation des centres anciens n'y est pas non plus étranger. Cela rejoint les préoccupations que notre commission exprime depuis un certain nombre d'années. Parmi les bonnes nouvelles

J'ai le plaisir d'appartenir à une région, le Grand Est, qui le fait déjà ; comme je suis conseiller régional, je m'occupe évidemment des questions de patrimoine, là-bas comme ici. Enfin, grande nouvelle- nous attendons avec impatience le collectif budgétaire -, le loto du patrimoine est créé. J'ai le souvenir que, voilà un certain nombre

Ces nouvelles ressources seront particulièrement nécessaires, parce que les crédits d'entretien et de restauration sont, chaque année, insuffisants par rapport aux besoins, et ce de manière structurelle. La mission de recensement du patrimoine en péril, que le

du nom du premier inspecteur général des monuments historiques ; cette base constitue un inventaire complet des besoins. La suppression de la réserve parlementaire, que je ne peux pas empêcher d'évoquer, a fait malheureusement disparaître une ressource très utilisée par beaucoup de parlementaires pour aider les petites communes dans la restauration. Il est donc essentiel que les crédits puissent être rétablis d'une autre manière, pour aider tous les patrimoines, y compris d'ailleurs celui du XX siècle. J'ajoute que les propriétaires des monuments historiques doivent être soutenus aussi, car les difficultés s'amoncellent pour

attentifs aux décisions qui seront prises dans le cadre de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, que vous avez initiée et qui est nécessaire, car l'annualité budgétaire n'est guère compatible avec le financement du patrimoine. C'est pour ces raisons que je donne un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Patrimoines

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un contexte marqué par la nécessité de restaurer la cohésion sociale, le rôle de l'art et de la culture demeure essentiel.

culture du plus grand nombre et le développement de la vie culturelle de proximité. L'effort significatif réalisé en direction de l'éducation artistique et culturelle était réclamé depuis longtemps.

la question du maillage des territoires a une résonance particulière dans notre assemblée. Compte tenu de cet objectif, nous sommes un peu surpris et inquiets de la baisse des crédits, hors structures labellisées et hors réseau, qui pourrait mettre en danger l'aménagement culturel équilibré des territoires, notamment dans les zones rurales. De manière générale, il est temps de faire des collectivités territoriales de véritables partenaires et même des coconstructeurs de la politique culturelle,

Aussi séduisante qu'elle puisse paraître de prime abord, cette idée comporte un certain nombre d'écueils dans lesquels il sera difficile de ne pas tomber ; l'expérience italienne, brandie par le Président de la République pour justifier sa proposition pendant la campagne, en constitue justement une illustration.

de donner un blanc-seing à un pass qui ne permettrait pas aux jeunes de diversifier leurs habitudes culturelles, qui remettrait en cause la diversité et qui, en définitive, créerait un effet d'aubaine pour les GAFA. Quant à son financement pour les années à venir, il suscite encore bien des interrogations ... Ce budget s'accompagne de fortes inflexions : l'accent en faveur de l'éducation artistique et culturelle, dont j'ai parlé, l'attention

Notre devoir de vigilance nous imposera d'en contrôler la mise en oeuvre, pour s'assurer que l'on ne dévie pas des objectifs fixés et que les résultats attendus sont bien au rendez-vous.

ministre, mes chers collègues, la mission « Culture » du projet de loi de finances pour 2018 présente des crédits de 2,9 milliards d'euros, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2017. Dans un contexte de réduction de la dépense publique, cette augmentation des crédits accordés à la culture mérite d'être saluée, et, tenant compte du rôle primordial des questions culturelles dans notre société comme vecteur de cohésion sociale objet de lutte contre les inégalités, notre groupe veut souligner cette initiative. Cette politique de soutien financier à la culture trouve aussi un écho dans le renforcement des crédits accordés aux directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. Celles-ci seront dotées, en 2018, d'un budget de 813 millions d'euros, en augmentation de 43 millions d'euros par rapport à 2017. Ce maillage culturel territorial et cette collaboration soutenue avec les collectivités territoriales sont plus qu'importantes. C'est en effet sur le terrain que ces projets culturels doivent être menés pour toucher le plus grand nombre de nos concitoyens évidemment, dans nos écoles, où nos élèves se forment chaque jour à la lecture et aux pratiques artistiques. L'augmentation du budget de l'éducation artistique et culturelle, pour atteindre 114 millions d'euros, soit une dotation supplémentaire de 35 millions d'euros en 2018, votre engagement conjoint avec M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, à défendre ces pratiques sont des marqueurs forts de notre volonté de croire en notre jeunesse et de lui donner les moyens de s'émanciper dans cette nouvelle société. Sur le programme 175 « Patrimoines », le budget devait répondre à de nombreux défis : l'étude des conclusions du rapport sur les musées au XXI siècle, le le projet d'année européenne du patrimoine, la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour l'architecture, etc. Ces défis nous semblent relevés. En revanche, notre collègue Philippe Nachbar, vous a alertée, en réunion de commission, sur le problème de la sous-consommation des crédits de l'action Patrimoine monumental de ce programme. Nous espérons que vous pourrez rapidement y apporter des solutions. Par ailleurs, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, notre groupe, comme Mme la présidente de la commission de la culture, avait proposé d'exonérer d'impôt sur la fortune immobilière les monuments historiques ouverts au public, sous condition d'une détention d'au moins quinze Notre patrimoine est « en péril ». Même si le mot est fort, il n'en demeure pas moins que nos monuments ont besoin d'être régulièrement entretenus. Si nous n'agissons pas, ce sont des pans entiers de notre histoire qui disparaîtront. Le fait que 12 millions de Français se soient déplacés à l'occasion des Journées du Patrimoine prouve bien tout l'intérêt de nos concitoyens pour notre histoire. La création d'un fonds de soutien à la restauration du patrimoine protégé en milieu rural, doté de 15 millions d'euros, nous paraît aller dans le bon sens, et nous étudierons avec attention les propositions à venir de la mission conduite par Stéphane Bern sur le patrimoine en péril. Sur les programmes 131, « Création », et 224, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

et nous espérons que la réunion de l'ensemble des acteurs concernés- acteurs publics et privés, élus, responsables de la vie culturelle et jeunes -permettra de donner à ce dispositif toutes ses chances de réussite. Deux autres Deux autres sujets me semblent importants pour la poursuite des débats. Ils nous ont d'ailleurs conduits à déposer des amendements. Le premier concerne le financement du Bureau export de la musique française. L'Assemblée nationale a déjà voté une augmentation des crédits de cet outil important de rayonnement international de la scène française. Nous avons souhaité lui emboîter le pas pour aller plus loin et pouvoir ainsi faire concurrence aux géants anglo-saxons. Le second amendement vise à revaloriser la subvention du ministère de la culture à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Celle-ci connaît depuis plusieurs années un fort déficit structurel en raison de nombreuses contraintes financières. Nous avons souhaité l'accompagner.

cette sanctuarisation est déjà un signal encourageant. La culture, dans son ensemble, sera pérennisée en 2018. Tout en étant d'un naturel optimiste, je reste prudente, car je m'interroge : ces moyens seront-ils suffisants pour insuffler une dynamique de transformation ? Si l'on s'attache à l'évolution des crédits budgétaires ligne par ligne, mon analyse est plus nuancée. Pour commencer, je tiens à relever la volonté de développer l'éducation artistique et culturelle. Le bien-fondé de l'effort budgétaire porté sur le financement de ces actions n'est plus à démontrer. C'est un outil très efficace pour démocratiser l'accès de tous les enfants à la culture. Les membres du groupe du RDSE et moi-même saluons cette orientation, qui sera très utile pour lutter contre les fractures culturelles et progresser vers l'égalité d'accès de tous à la culture. C'est en effet sur les bancs de l'école et dès le plus jeune âge que cela se joue. néanmoins souhaité qu'un budget plus important y soit consacré, dès maintenant. Pour moi, cette dépense aurait dû être prioritaire par rapport au pass culture. En effet, si je suis convaincue du bien-fondé de ce sésame, je serai vigilante sur les conditions de sa mise en oeuvre, car beaucoup de questions d'ordre pragmatique se posent. se posent. Il me semble important de tenir compte des expérimentations qui se déroulent déjà sur notre territoire et de bien définir les conditions dans lesquelles les jeunes pourront bénéficier de ce dispositif. Si l'on ne leur offre aucune préparation ou aucun accompagnement dans leurs choix, je doute que le résultat soit à la hauteur de nos ambitions. Il est donc urgent de prendre du temps pour encadrer ce dispositif, comme l'a précisé notre collègue Sylvie Robert. Je ne perds néanmoins pas de vue que ces crédits contribueront indirectement à redynamiser la demande auprès des artistes et du secteur de la création artistique et culturelle dans son ensemble. pour citer les paroles de l'acteur Philippe Torreton, « la culture est une force de frappe économique » ; comme lui, j'en suis persuadée. Concernant l'augmentation de 3 millions d'euros des crédits alloués au plan Conservatoires, ce nom est presque une tromperie Il s'agit plutôt d'un plan Chorales, qui bénéficiera non pas directement aux conservatoires, mais bien aux établissements scolaires. Nous pouvions là aussi espérer davantage de progrès dans la mise en oeuvre des réformes prévues par la loi LCAP.

pu bénéficier de deux rapports, celui de M. Malvy et celui de M. Dauge, qui ont permis de lancer des pistes de travail pour mieux valoriser le patrimoine de nos territoires. Des expérimentations sont lancées dans trois régions pilotes pour évaluer la mise en oeuvre des recommandations faites en vue de revitaliser les petites communes, les centres-villes et les villes moyennes. Il reste à espérer que les expérimentations réussies seront étendues au reste de notre territoire. En outre, une aide de 15 millions d'euros, transitant par les DRAC, est prévue pour aider les petites communes à faible potentiel financier à sauvegarder leur patrimoine historique.

et que, d'autre part, le secteur culturel dans son ensemble s'inquiète de l'annonce de l'arrêt des contrats aidés. Pourquoi procéder maintenant à cette coupe massive dans les crédits destinés à soutenir l'emploi dans le spectacle, avant même d'avoir évalué les premières mesures en question et essayé de les améliorer ? mon propos en rappelant que les mesures de sécurité sont désormais devenues une dépense incontournable pour l'organisation de tout événement artistique et culturel. Nous devons prendre en compte cet état de fait dans la programmation budgétaire. En effet, il est à craindre que le budget consacré aux mesures de sécurité n'empiète sur celui de la création. Je pense, par exemple, à l'organisation de festivals dans nos départements et nos régions. ce qui est ressorti de l'enquête réalisée auprès des sénateurs membres du groupe de travail sur les arts de la scène, de la rue et des festivals en régions, que je préside. Cette question est d'autant plus importante que le fonds d'urgence créé en décembre 2015 s'arrêtera à la Madame la ministre, que pouvez-vous nous dire au sujet des crédits attribués au fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est censé s'y substituer ?

Monsieur le président, madame la ministre, cher collègue, j'aimerais commencer mon propos par une citation ; c'est une façon personnelle de rendre hommage à Jack Ralite, qui les aimait tant. Dans ses, Madeleine de Puisieux écrivait : « Il y a plus d'habilité à se tirer bien d'une aventure délicate qu'à l'entreprendre ; presque tous les commencements sont beaux, les milieux fatigants et les fins pitoyables. Il est rare qu'on finisse bien ce qu'on a commencé ; soit faute de lumière, soit faute de courage, on finit mal. Il y aurait un moyen d'arranger tout : ce serait de ne point commencer ou de ne jamais finir. Je vous souhaite donc, madame la ministre, beaucoup de courage pour retenir votre ministère dans la pente fatale vers laquelle l'entraînent des financiers zélés et lui éviter ainsi le dernier stade décrit par Madeleine de Puisieux. Il faut en effet toute l'habilité de vos services budgétaires pour nous expliquer que le budget est « en légère augmentation », alors que les crédits alloués à la culture passeront sous la barre symbolique de 1 % du budget de l'État, à périmètre constant. Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances ont clairement établi que c'est le rattachement extraordinaire à la mission du compte d'affectation spéciale « Pensions » qui permet de sauver les apparences et d'afficher cette pseudo-stabilité. Réduit à la seule mission « Culture », votre budget ne représente plus que 0,84 % de celui de l'État. M. Bruno Le Maire a fixé le cap en imposant « trois points de dépense publique en moins », et votre ministère n'échappe malheureusement pas à cet effort de contraction. Cette baisse des apports de l'État s'ajoute à celle des dotations aux collectivités, qui contribuent pour les deux tiers aux dépenses culturelles dans les territoires. Elles sont à la fois destructrices pour l'infrastructure culturelle et économiquement absurdes, car les dépenses culturelles ont un fort effet de levier et participent efficacement aux politiques de redynamisation des territoires, à la condition qu'elles s'intègrent dans une démarche globale. Dois-je rappeler que la contribution de la culture à l'économie française représente 3,2 % du PIB ? Avec un budget en réduction, vous avez donc choisi de définir des priorités pour tenter de mobiliser des moyens en leur faveur. ces priorités, ainsi que l'avait annoncé le Président de la République dans son discours de la Pnyx, prononcé quelques mois avant le lancement de l'année européenne du patrimoine Néanmoins, les mesures nouvelles que vous annoncez dans ce domaine sont financées par un redéploiement sévère au sein d'une enveloppe qui est, elle aussi, en baisse. Cette mobilisation se fait surtout aux dépens du patrimoine des musées et des archives. Ces institutions subissent une ponction sévère qui nous préoccupe au plus haut point. La situation financière des musées a été particulièrement affectée par la baisse de fréquentation consécutive aux attentats. Le nombre d'entrées n'a toujours pas retrouvé son niveau antérieur à cette crise ; la diminution des recettes a eu quant à elle des conséquences fâcheuses sur l'accueil des visiteurs, dont l'insatisfaction a augmenté. Les restrictions budgétaires vont surtout toucher les petites structures qui ne bénéficient pas d'apports extérieurs. Enfin, votre budget, comme de nombreux autres avant lui, consacre l'abandon par l'État de toute politique volontariste en matière d'acquisition. S'agissant du patrimoine monumental, qui constitue pourtant l'une des priorités déclarées de ce projet de budget, nous nous inquiétons de la baisse de 1,5 million d'euros des crédits de paiement. Cette baisse s'ajoute, pour l'ensemble du ministère, à une prévision de consommation de crédits de paiement pour des autorisations d'engagement antérieures qui s'élève à plus de 227 millions d'euros, soit 25 % des crédits de paiement du présent projet Ce rapport considérable est la conséquence de la difficulté chronique qu'éprouvent les services déconcentrés à monter des dossiers et consommer les crédits. Force est de reconnaître que les capacités du ministère de la culture à programmer ou achever de grandes opérations de restauration du patrimoine sont devenues très limitées. Cette impéritie est d'autant plus inquiétante qu'elle concerne des biens prestigieux du Centre des monuments nationaux comme le Panthéon, le château de Pierrefonds, les remparts de la cité de Carcassonne ou- faute politique quand on vient présenter un budget au Sénat -les décors du château de Rambouillet. Ces faibles capacités d'investissement ne laissent pas d'inquiéter alors que ce ministère aura à conduire, dans les prochaines années, plusieurs lourdes opérations immobilières autour du Grand Palais, de la Cité du théâtre, du Centre national des arts plastiques ou du château autre sujet d'inquiétude : la baisse du plafond d'emploi, alors même que celui fixé par le budget pour 2017 n'a pas été exécuté. Cette fragilisation des moyens humains de votre ministère, qui touche surtout vos services déconcentrés, risque de compromettre gravement la mise en oeuvre de votre politique de partenariat avec les collectivités. Je pense plus particulièrement au mécanisme partenarial et incitatif d'aide à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales à faible potentiel financier, qui est pourtant l'une des priorités de ce projet de budget. Plus généralement, la baisse continue des moyens humains de votre ministère et de ses opérateurs aura des conséquences graves et irrémédiables sur l'action et l'offre culturelles : des musées et des monuments vont fermer, les collectivités vont perdre des interlocuteurs précieux. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, nous voterons contre ce projet de budget, qui est en contradiction avec les objectifs politiques de votre ministère. La parole est à Mme Sonia de la Provôté. Monsieur le

l'évolution globale des crédits dévolus à la culture est rassurante. Je ne m'étendrai donc pas longuement sur le sujet, qui a été bien présenté par nos rapporteurs, dont je salue au passage l'excellence du travail.

C'est une bonne chose, car le monde de la culture, dans son ensemble, a besoin de cet équilibre. J'appuierai donc mon propos sur les sujets particuliers qui nous interrogent. Le premier sujet, vous vous en doutez, est le pass culture, qui mérite que l'on s'y attarde.

Ces 5 premiers millions sont destinés à la consultation des jeunes, à la recherche de partenaires, à la mise au point d'une application et à des expérimentations prévues en fin d'année.

qui ne donnerait accès qu'à une culture strictement calquée sur les goûts et appétences habituels du jeune ; on connaît la puissance des algorithmes individuels et l'usage dévoyé qui en est fait en la matière. souhait est bien que le jeune puisse accéder à une offre culturelle différente, moins spontanément attractive, mais source d'un enrichissement culturel et personnel à coup sûr bien meilleur. Autrement dit, l'objectif est bien celui d'un accès à d'autres propositions que celles qui inondent le marché privé de la culture, qui est dominé, notamment, par les offres des GAFA. Cet objectif, en réalité, est majeur. Si l'on y parvient, ce sera un puissant soutien de la diversité culturelle.

Cela pose la question d'une politique très construite articulant la culture et l'éducation. Les deux ministères ont d'ailleurs fait savoir qu'ils souhaitaient travailler ensemble. Par-delà l'affichage, il faudra expliciter quels moyens financiers et humains seront mutualisés aussi clarifier les moyens et les outils pédagogiques et de médiation qui seront mis en oeuvre en fonction de l'âge et du parcours de l'enfant, puis du jeune. Le second sujet sur lequel je souhaitais appeler à la vigilance est celui des conservatoires.

La hausse budgétaire devient ainsi toute relative. Nous ne sommes pas opposés, bien au contraire, au plan Chorales ; c'est même une bonne idée. Néanmoins, la question du recentrage des conservatoires sur leur vocation première, à savoir l'enseignement artistique, doit être posée ici avec fermeté. Il est nécessaire de réaffirmer la vocation de ces lieux, qui sont des références, d'où partent les formateurs et où se construit l'excellence ; c'est leur rôle. Le risque est la dispersion des missions des conservatoires, qui n'auront pas les moyens de tout faire. Il faudra veiller à ce que leur coeur de métier soit préservé. leurs missions premières reste extrêmement contraint. La part étatique du financement des conservatoires atteindra cette année 20 millions d'euros. Elle était de 35 millions

En attendant, la réalité oblige les conservatoires à être principalement financés par les collectivités. Or celles-ci ne pourront pas pallier les besoins supplémentaires.

la création. La priorité donnée à la vie culturelle dans les territoires et le renforcement des aides à la diffusion des oeuvres est une bonne chose, car la diffusion est assez souvent ce qui fait défaut dans les territoires. Néanmoins, ce choix ainsi que l'orientation renforcée vers les labels appellent à une certaine vigilance en ce qui concerne la création et l'accompagnement des artistes. En effet, si l'on veut maintenir ce qu'on appelle « l'effervescence culturelle », ce qui fait la vitalité de la vie artistique dans tous les territoires, il faudra pallier la baisse des moyens des collectivités territoriales, dont les arbitrages en matière culturelle deviennent de plus en plus difficiles. En outre, la disparition des emplois aidés, nombreux dans les structures culturelles, est un élément supplémentaire de fragilisation, par exemple pour le spectacle vivant. Il vigilance, car la diversité et la liberté culturelles sont un combat plus qu'actuel, surtout face au risque porté par de grands groupes qui concentrent l'offre et proposent de plus en plus une culture uniformisée.

la réussite des grands musées, qui sont parvenus à diversifier leurs ressources. Pour autant, rien n'est jamais inscrit dans le marbre, et les efforts consentis ne doivent pas occulter les besoins à venir. second lieu, nous nous réjouissons qu'une part des gains de la Française des jeux finance enfin le patrimoine, même si la fourchette reste large : 5 millions ou 20 millions d'euros, ce n'est pas tout à fait la même chose ! Il est pertinent d'avoir fléché cette participation vers la Fondation du patrimoine, dont le système est souple et réactif, et l'implantation territoriale performante. Ce sera particulièrement utile pour la protection du patrimoine non classé, patrimoine vernaculaire présent surtout dans les communes rurales : les églises, les halles, les lavoirs ou encore les granges. C'est tout ce qui appartient à notre mémoire collective. Les besoins sont grands.

Je pense que le patrimoine de la reconstruction, qui concerne beaucoup de centres-villes et centres-bourgs, méritera d'être, pour une grande part, sauvegardé. Ce qui fait patrimoine relève de grands ensembles urbains, ce qui implique des coûts. On ouvre ici tout un pan de la dépense publique et de l'accompagnement de l'État, qui peut prendre des dimensions majeures.

La réflexion sur les moyens est d'autant plus urgente que, pour l'heure, rien ne semble devoir remplacer la disparition de la réserve parlementaire et le rétrécissement des financements des conseils départementaux, appelés eux aussi à des arbitrages budgétaires de plus en plus complexes. Pour les petites communes, cela s'avère particulièrement vital. On peut donc se réjouir de la préservation globale des crédits du patrimoine et, encore plus, de la création d'un fonds incitatif, doté de 15 millions d'euros, réservé aux collectivités territoriales à faibles ressources financières, même si nous estimons dès à présent que ce fonds sera probablement insuffisant. le groupe Union Centriste soutient les orientations financières globales du présent budget, mais il attend que, dès 2018 et dans le cadre du budget pour 2019, des clarifications soient apportées sur le pass culture, sur le devenir et l'accompagnement de la création, sur le soutien aux artistes, sur la proposition d'un véritable plan Conservatoires et, enfin, sur le suivi et l'adéquation des moyens mis en oeuvre pour la préservation

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « Presque tout ce qui caractérise l'humanité se résume par le mot culture », affirmait François Jacob. Vecteur de tolérance, d'émancipation et d'épanouissement, elle est tout à la fois porteuse de diversité dans les formes qu'elle revêt et gage d'unicité et de cohésion en ce qu'elle favorise les échanges et le partage, ce qui permet de « faire société ». Sans culture, point d'humanité : tel était le message de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui établissait celle-ci comme un droit fondamental. À l'aune d'un tel constat, l'enjeu du budget alloué pour 2018 à la culture apparaît primordial. Nous nous félicitons, madame la ministre, que vous nous soumettiez un budget conforté. Cette légère hausse globale masque toutefois une certaine modification des équilibres internes le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation culturelle » bénéficie d'un effort plus important, tandis que les crédits du patrimoine sont en baisse. Nous nous réjouissons de la priorité donnée à la jeunesse et à l'accessibilité de toutes et tous à la culture. Une véritable coopération entre le ministère de l'éducation nationale et le vôtre est attendue depuis de nombreuses années ; elle semble commencer, mais à hauteur de 3 millions d'euros seulement ! Pourtant, face à cette priorité affichée d'une démocratisation culturelle effective dans l'ensemble des territoires, certaines dispositions inquiètent les acteurs culturels et les élus. En tant que compétence partagée, la politique culturelle doit faire l'objet d'une réelle collaboration entre l'État et l'ensemble des collectivités. Ces dernières investissent à hauteur de 57 %, et le Gouvernement se doit d'encourager leurs actions, garantes d'un développement de l'offre culturelle en tout point du territoire. Toutefois, à l'heure des budgets serrés, la culture constitue encore trop souvent la variable d'ajustement. Le risque qui en découle est bien celui d'une véritable fracture territoriale. J'ai une autre inquiétude : l'annonce de la suppression des contrats aidés, qui constituent une part non négligeable des emplois

à destination de publics multiples et, notamment, des plus fragiles. Sans les contrats aidés, ces structures se trouvent bouleversées. Cela va à rebours d'un accès équitable à la culture. Ces contrats aidés, très souvent pérennisés, pour de nombreux jeunes artistes une première insertion dans la vie professionnelle en lien avec leur pratique. Les crédits du FONPEPS, dont le budget- j'insiste sur ce point -a été réduit de moitié, ne doivent pas constituer une solution d'urgence pour remplacer ces contrats aidés supprimés. Vous avez marqué votre volonté de soutenir les artistes dans leurs conditions de vie, artistes sans lesquels toute politique culturelle serait vaine. Un effort budgétaire plus important pourrait être consenti afin de favoriser leur accompagnement vers la vie active : aujourd'hui, seuls 10 % des élèves diplômés parviennent à vivre exclusivement de leur pratique artistique, faute de moyens et d'accompagnement. Une telle déperdition de talents est extrêmement dommageable. Notre rapporteur pour avis Sylvie Robert a évoqué la question des écoles d'art, que nous envient beaucoup de pays. La démocratisation culturelle et l'attention portée à la transmission des savoirs passent aussi par un nécessaire soutien à ces écoles et à leurs personnels. Par ailleurs, je souhaiterais évoquer le mécénat culturel. S'il n'est pas question de le remettre en cause, il ne doit pas constituer un prétexte au désengagement financier de l'État. En effet, le mécénat des grands groupes comme celui des multinationales concerne surtout les grandes villes et peu les territoires ruraux : il s'agit là d'un autre point de vigilance, car il ne doit pas constituer une nouvelle fracture entre territoires. Le budget dédié à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes est transversal et concerne tous les ministères, mais le vôtre, madame doit en être le porte-voix tant l'image que la culture française véhicule dans le monde est emblématique de notre société.

d'abord de reconnaître l'effort accompli en faveur de la culture, en particulier en faveur de la mission « Culture », dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. En effet, s'agissant des crédits budgétaires sur lesquels s'exerce le contrôle de la représentation nationale, le budget global pour 2018 du ministère de la culture est relativement stable, voire en légère augmentation- selon les interprétations là où 58 % des communes françaises ont été contraintes de réduire la voilure. Au-delà des questions budgétaires, notre groupe partage votre vision, madame la ministre, qui fait de la culture l'un des fondements de l'éducation. À cet égard, je salue votre volonté et celle de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de faire davantage entrer la culture à l'école, qui est le lieu privilégié pour permettre à tous, notamment à ceux qui en sont le plus éloignés, d'accéder à l'éducation artistique et culturelle. C'est la raison principale pour laquelle le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission « Culture ». Si cette relative stabilité est à souligner, l'évolution des équilibres internes au budget soulève toutefois nombre d'interrogations et d'inquiétudes. Le travail en profondeur de la commission de la culture, dont je salue la bienveillante présidence de Catherine Morin-Desailly, a d'ailleurs suscité de nombreux débats, extrêmement intéressants et passionnés, dans lesquels, par-delà nos sensibilités diverses, nous avons dû constamment tenter de démêler ce qui pouvait relever de l'effet d'annonce ou d'une réalité crédible. Prenons par exemple le point fort de ce budget, qui est sans aucun doute l'effort qu'il assume en direction des territoires. vrai que les crédits déconcentrés en faveur des collectivités et des citoyens sont en hausse de 6 %, à 860 millions d'euros, ce dont nous nous félicitons. En vérité et dans le détail, si vous souhaitez véritablement aider les petites collectivités rurales à entretenir leur patrimoine historique avec un fonds dédié à hauteur de 15 millions d'euros seulement, j'ai bien peur que ne vous soyez loin du compte, surtout lorsque l'on connaît, parce que l'on a été élu local, le coût monstrueux de la moindre reprise en sous-oeuvre d'un bâtiment, si tant est que la DRAC ait daigné vous donner préalablement une autorisation dans les délais impartis ... Si l'on ajoute à cette situation préoccupante la suppression de la réserve parlementaire, qui permettait de venir en appui des nombreuses demandes, de graves difficultés sont en vue, comme l'a souligné Philippe Nachbar, parce que Nachbar, parce que la politique patrimoniale dépasse le simple cadre culturel. Elle contribue à réduire la fracture territoriale et recrée de l'attractivité économique ou touristique dans des communes, souvent rurales, qui possèdent un patrimoine. Entretenir ce patrimoine et rénover les centres historiques dégradés est donc une absolue nécessité. Nous avons par ailleurs d'autres interrogations. Comment ne pas être favorable à la rentrée scolaire en musique et au plan Chorales, sachant combien la musique peut apporter à notre jeunesse ? Je suis bien placé pour en parler ... Comment ne pas être tout autant favorable à l'ouverture des bibliothèques le dimanche ? ? Là encore, les moyens réels sont-ils à la hauteur de l'ambition collective ? Nous en doutons ! Aujourd'hui, ce sont des communes exsangues et sans cesse montrées du doigt comme dépensières qui doivent pourtant financer, sur leur budget de fonctionnement, des musiciens intervenants ou des personnels du secteur culturel. Certes, vous avez confié, au mois de septembre dernier, une mission à l'académicien Érik Orsenna et les évaluations sont en cours, mais, encore une fois, aucun budget spécifique n'est prévu. Au titre des satisfactions, je tiens à saluer, madame la ministre, votre annonce du principe de compensation de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs, qui contribuent activement au dynamisme et au rayonnement culturel de notre pays. C'était une préoccupation de notre groupe, et je me félicite qu'elle ait été entendue par le Gouvernement. Il est en effet vital que les écrivains, les compositeurs, les photographes, les traducteurs, les sculpteurs, qui vivent des droits d'auteur et qui ne cotisent pas à l'assurance chômage, ne subissent pas l'impact d'une hausse de la CSG, alors même qu'ils contribuent activement au dynamisme et au rayonnement culturel de notre pays. Malheureusement, au-delà de certains motifs de satisfaction, des sujets d'inquiétude, déjà évoqués en commission, demeurent. Il me paraît essentiel d'en rappeler ici quelques-uns. au financement des travaux du Grand Palais ou d'autres grands chantiers patrimoniaux, sans parler de l'état de délabrement du palais Garnier qui pose question. Je pense aussi à la baisse des autorisations d'engagement des crédits consacrés aux musées la fin du mécanisme de soutien à la sécurisation des salles de spectacle. Je pense également au manque de reconnaissance des enseignants des écoles d'art régionales, à la baisse des crédits alloués à la Philharmonie, qui, à travers ses trente orchestres du Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale,

Le Gouvernement veut donner à chaque jeune de dix-huit ans un pass de 500 euros destiné à financer des entrées dans des musées ou des monuments historiques, des places de spectacle, des livres ou de la musique. Soit La mission chiffre le coût final à l40 millions d'euros, alors que son périmètre n'est pas encore calé. Son coût pourrait, en réalité, se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros. En outre, les milieux culturels s'inquiètent, à juste titre, du fait que ce pass puisse générer un effet d'aubaine pour les géants internationaux qui ne financent pas la culture en France, comme Netflix et Amazon, sans parler des risques de détournements frauduleux observés par exemple en Italie, où cette mesure a déjà été tentée. Par ailleurs, même si tout le monde a bien compris que le jacobinisme a la vie dure, il eût été il eût été certainement utile d'observer attentivement et d'analyser préalablement ce qu'il se fait déjà dans certaines régions françaises, notamment en Pays de la Loire, région chère au président de notre groupe, Bruno Retailleau, où ce type de dispositif existe depuis bientôt vingt ans. Les expérimentations et initiatives locales sont autant de laboratoires qui font la richesse de notre pays. Les ignorer, même si c'est la mode, est une erreur, et le Sénat est dans le rôle de représentant du territoire que lui confère l'article 24 de la Constitution lorsqu'il le rappelle. Comment ne pas sourire lorsqu'un présentateur, ô combien médiatique, réussit à obtenir en un clin d'oeil le désormais fameux loto du patrimoine, alors que des sénateurs, certes moins médiatiques mais d'une compétence avérée, le recommandaient depuis des années sans avoir plus de chances au grattage qu'au tirage Alors, oui, madame la ministre, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission « Culture », mais gardera un oeil particulièrement attentif sur l'exécution budgétaire ainsi qu'une oreille avisée sur l'harmonie de l'ensemble.

consolidé de la mission « Culture » témoigne de l'importance accordée par le Président de la République à l'implication de l'État dans ce domaine et, plus généralement, au rôle joué par la culture comme facteur de cohésion sociale et d'agrégateur constructif de nos identités collectives. Pour mémoire, on rappellera combien cette mission avait vu ses moyens singulièrement diminuer durant les trois premières années du précédent quinquennat, avant de reprendre par la suite un peu de couleurs, sans parvenir toutefois à les ramener au niveau de 2011. pour un premier exercice budgétaire de la nouvelle majorité présidentielle, cette consolidation est de bon augure, d'autant que le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit une augmentation de 50 millions d'euros au cours des trois années à venir. « consolidation » ne signifie heureusement pas ici « reproduction à l'identique » des choix passés. Cela reviendrait en effet à une forme de conservatisme culturel tout le contraire de ce dont le secteur a besoin aujourd'hui. Au cours des décennies écoulées, les pratiques culturelles des Français ont considérablement évolué. L'explosion du numérique et son impact sur celles-ci constituent l'un des exemples les plus visibles de ce bouleversement, mais ce n'est pas le seul. Face à ces changements, nos politiques publiques sont restées beaucoup trop statiques et pas toujours à la hauteur des défis à affronter. C'est le revers de la création, en 1959, d'un grand ministère des affaires culturelles en France. L'institutionnalisation à la française a rarement été source d'agilité et de réactivité ... Parmi les quatre grandes missions historiques assignées à ce ministère- encourager la création, protéger et valoriser notre patrimoine, assurer le rayonnement international de la culture française et démocratiser l'accès de nos concitoyens à la culture -, cette dernière, qui est pourtant la légitimation première de toute politique publique dans un État démocratique digne de ce nom reste pourtant pourtant sur un échec patent. « La culture pour tous » est en effet loin d'être une réalité dans notre pays. La dernière grande étude conduite par le ministère sur les pratiques culturelles, qui date de près de dix ans, ans, souligne que 52 % de nos concitoyens ont une fréquentation nulle ou très exceptionnelle des équipements culturels. Certes, nos grands établissements culturels- en particulier les musées -enregistrent des niveaux élevés de fréquentation, mais leur clientèle est de plus en plus touristique et étrangère. Durant le dernier quinquennat, les ministres de la culture qui se sont succédé ont, de façon un peu malhabile, tenté de justifier les moyens qui leur étaient alloués par un discours de nature toujours plus économique- attractivité touristique du pays, nombre d'emplois induits, retombées économiques du secteur reléguant de fait la démocratisation de la culture au rang d'objectif louable, mais non prioritaire ... Au mois de mai dernier dans les colonnes du, Michel Guerrin posait crûment cette question Comment séduire les 50 % de Français exclus de la culture ? Disons-le brutalement, la culture est le seul secteur où les pauvres paient des impôts qui contribuent à construire une offre qui ne profite qu'aux riches. Il poursuivait en rappelant que le problème de l'accès à la culture se pose non seulement en termes d'inégalités sociales, mais également en termes géographiques : « Nos flambeaux culturels sont plantés dans les grandes villes et, plus que cela, au centre de ces métropoles : le déséquilibre entre territoires est vertigineux. » Dans un rapport de 2004, trop prestement passé aux oubliettes, Bernard Latarjet pointait déjà un inquiétant paradoxe : le nombre d'artistes et de spectacles ne cesse d'augmenter depuis trente ans, alors que le public de l'offre culturelle stagne. C'est bien pour cette raison que que le Président de la République a choisi de faire de l'accès à la culture sa priorité. À quoi servent en effet une politique de soutien à la création, une politique de préservation et d'enrichissement du patrimoine national, une politique d'acquisitions d'oeuvres et d'édification de nouveaux établissements, si celles-ci ne sont pas accompagnées d'une vigoureuse politique de diffusion et d'accessibilité sur tout le territoire national et d'un réel effort à destination de l'ensemble du corps social et plus seulement d'une petite élite culturelle ? À quoi cela sert-il si nous ne savons pas nous adapter aux nouvelles pratiques culturelles de la jeunesse de mieux leur transmettre notre richesse artistique et patrimoniale en pleine intelligence et complémentarité avec les moyens déployés par notre système éducatif ? Cette volonté politique d'affronter enfin le défi de l'accessibilité de la culture de qualité au plus grand nombre, c'est celle qui, dans cette mission budgétaire, s'incarne notamment à travers une augmentation très sensible des crédits de soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle : 173 millions d'euros en 2018, contre 119 millions Faire davantage circuler sur tout le territoire les grandes oeuvres que recèlent nos musées parisiens, faire tourner en France les spectacles mis en scène par nos grands théâtres nationaux, élargir encore les horaires d'ouverture de nos bibliothèques et de nos musées et- plus qu'une cerise sur le gâteau -préfigurer la mise en place d'un pass culture destiné à notre jeunesse, en prenant au préalable soin de dresser un véritable état des politiques tarifaires existantes, de bien circonscrire les champs culturels concernés pour mieux calibrer cette offre et les moyens pour la faire connaître afin de la rendre effective et performante dès le courant de l'année 2019, c'est bien cela dont la mission « culture » pour 2018 est le nom. L'enjeu est de taille. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, c'est sans réserve que le groupe La République En Marche votera les crédits de cette mission. La parole

Derrière une volonté affichée de faire du patrimoine un axe majeur de votre politique culturelle, madame la ministre, ces chiffres nous alertent sur la réalité des moyens budgétaires que le Gouvernement a souhaité accorder à ce programme, qui demeure le parent pauvre de votre budget. C'est le seul programme de la mission qui ne bénéficie pas d'une augmentation, alors que la transmission du patrimoine aux générations futures constitue l'une de vos orientations stratégiques pour l'année à venir. Je rappelle pour mémoire que 2018 sera l'année européenne du patrimoine.

de leurs habitants et de leurs commerces, leurs patrimoines bâtis se dégradent. La politique patrimoniale est essentielle pour recréer de l'attractivité économique, mais aussi pour réduire la fracture territoriale entre les grandes métropoles et la France des petites villes et de la ruralité. C'est donc aussi un enjeu de cohésion sociale. Cette situation alarmante doit être renversée par une politique volontariste en mots, mais surtout en actes et sur la durée. Une revitalisation de grande ampleur est vitale pour la survie de ces territoires et de leurs centres historiques. La loi LCAP a permis des avancées importantes avec la création des sites patrimoniaux remarquables, qui permettent de recréer des conditions d'attractivité économique et touristique, dans ces communes. Le chantier est immense, et il faut aller plus loin. Nous nous réjouissons des quelques mesures que le Gouvernement propose pour la revitalisation de ces territoires. Je pense au fonds de 15 millions d'euros pour la restauration du patrimoine situé dans les communes de moins de 10 000 habitants ou aux 9 millions d'euros concernant la revitalisation des centres-bourgs et des petites villes. Nous ne pouvons que vous encourager en ce sens. Pour aller plus loin, je compte proposer des amendements visant à faire bénéficier ces territoires fragilisés d'une fiscalité plus incitative. J'en viens aux autres points du programme. Nous nous inquiétons des baisses importantes sur plusieurs actions essentielles

le fonds du patrimoine, qui permet d'enrichir les collections des musées de France, passe de 3,6 millions d'euros en 2017 à 1,09 million d'euros en 2018. Les petits musées nationaux de province seront les premières victimes de ces coupes, madame la ministre. Où est donc la cohérence ? Ces dispositions sont en contradiction avec votre volonté de recréer de l'attractivité dans les petites villes et les centres anciens.

cogérés par l'État et les collectivités territoriales, qui remplacent petit à petit les dépôts archéologiques. Les CCE ont un rôle majeur en matière de conservation du patrimoine archéologique, dans le double but de favoriser la recherche et la vulgarisation des activités scientifiques de l'archéologie. Outre la plus grande accessibilité des objets issus des fouilles, ces structures sont nécessaires dans les territoires, tant pour valoriser l'histoire locale, qui constitue une forme importante de lien social, que pour contribuer à l'acceptabilité des recherches archéologiques, en particulier de l'archéologie préventive. Il s'agit donc à nouveau d'une coupe dans les moyens à destination des territoires. Je conclurai sur l'action n° 01, Patrimoine

Cette baisse des crédits est donc on ne peut plus inquiétante. Il faut conclure, chère collègue ! Faisons en sorte de ne pas nous engager dans le cercle vicieux de la dégradation et du manque d'entretien, qui aboutirait au scénario catastrophe où l'État serait contraint de vendre nombre de ses monuments historiques. L'action Patrimoine monumental sert trop souvent de variable d'ajustement pour financer d'autres actions. Pour conclure, madame la ministre, si plusieurs dispositions vont dans le bon sens, les crédits que vous accordez au programme « Patrimoines » ne nous paraissent pas à la hauteur des enjeux. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, sénateurs, en vous présentant aujourd'hui le premier budget de la culture de ce quinquennat, je vous présente bien plus que le budget d'un ministère : c'est une part essentielle du projet présidentiel et de la feuille de route du Gouvernement. Dans tout projet politique, l'ambition donnée à la culture est en effet l'un des miroirs les plus clairs du type de société que l'on souhaite porter. Presque tout ce qui caractérise l'humanité se résume par le mot culture », affirmait François Jacob, comme vous l'avez rappelé, madame Blondin. Notre ambition est majeure. Le Président de la République n'a cessé de le rappeler tout au long de sa campagne, et il l'a réaffirmé devant le Parlement réuni en Congrès : la culture est au coeur de son projet. Ce projet doit permettre à la France de relever les défis du XXI siècle pour rendre à notre pays son optimisme et pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. tel n'est pas le cas aujourd'hui. Comme vous l'avez souligné, monsieur Gattolin, nombre de nos concitoyens se sentent exclus, ou à contre-courant, des orientations prises, depuis quelques décennies : mondialisation, numérique, innovation, évolutions économiques et sociales, choix sociétaux. C'est d'abord pour tous ceux-là que je veux développer une politique culturelle : pour que tous ceux qui souffrent d'une forme d'exclusion, d'injustice ou de désoeuvrement puissent participer à la vie culturelle de leur commune, de leur région, de notre pays. Pour que tous ceux qui se disent que cette société avance sans eux, ou contre eux, aient accès à ce levier essentiel d'émancipation : l'exploration culturelle, la découverte d'un lieu, l'apprentissage d'un art. Notre politique culturelle doit être une politique d'émancipation pour chacun et de solidarité entre tous. En effet, la culture est ce qui, individuellement, nous tient le plus solidement debout et ce qui, collectivement, nous tient le plus solidement ensemble. pour que la culture joue ce double rôle, il faut combattre les logiques d'exclusion ou d'auto-exclusion qui la traversent elle-même. Tous nos citoyens ont accès à une forme de culture, mais, notre vrai défi, c'est l'exploration, la diversité. Des barrières et des déterminismes contraignent des millions de citoyens dans leurs choix culturels. Nous devons les faire tomber. C'est ici ma mission. Je me battrai- j'insiste sur

l'élan singulier que chacun dans cet hémicycle a sans doute un jour éprouvé. Pour cela, j'ai pris un parti clair : la politique culturelle que je promeus est une politique culturelle de proximité. Nous irons au-devant de ceux que ce ministère n'a pas réussi à toucher, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, dans les villes moyennes, en outre-mer et dans les quartiers prioritaires de la Nous donnerons à chaque citoyen les moyens de son autonomie. Le projet de budget pour 2018 en est la traduction directe. Les crédits de la mission « Culture » seront renforcés : ils s'établiront à plus de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 42 millions d'euros par rapport à 2017. Les moyens seront rééquilibrés en faveur des territoires. Les crédits déconcentrés seront en effet portés à 860 millions d'euros,

les associations. Madame Robert, nous coopérerons encore plus étroitement avec les collectivités territoriales : j'ai proposé aux associations d'élus de bâtir pour cela un nouveau cadre de contractualisation plus souple et plus solidaire. Nous innoverons en poussant ce ministère à agir aussi, beaucoup plus, en dehors de ses propres canaux institutionnels. Enfin, nous nous appuierons sur quatre relais privilégiés. Le premier Pour que la culture soit un levier d'émancipation pour chaque citoyen, elle doit occuper une place structurante dans le développement de chaque enfant. Nous allons la mettre au coeur du nouveau modèle d'école bâti par ce gouvernement. C'est une ambition que je partage avec Jean-Michel Blanquer,

de la maternelle au lycée. Le budget de l'éducation artistique et culturelle augmentera significativement dès l'année prochaine : il dépassera 110 millions d'euros, en hausse de plus de 30 millions d'euros.

Pour développer la pratique artistique, nous généraliserons à court terme un outil simple et concret : les chorales. Je m'exprimerai prochainement, avec le ministre de l'éducation nationale, sur la mise en oeuvre d'un plan Chorales. Les partenariats entre les écoles et les conservatoires sont féconds, je l'ai constaté récemment encore lors de mon déplacement à Rouen à vos côtés, madame la présidente de la commission de la culture. Je souhaite aussi qu'une Fête de la musique à l'école voie le jour, dont la première édition aura lieu le 21 juin nous développerons dès l'année prochaine les jumelages entre établissements scolaires et établissements culturels locaux : nos structures labellisées, les structures soutenues par les collectivités, comme les conservatoires, et les lieux patrimoniaux. L'objectif est d'avoir 100 % d'écoles jumelées d'ici à 2022, pour favoriser les sorties et les activités culturelles. Évidemment, nous soutiendrons aussi toutes les actions entreprises hors temps scolaire. Monsieur le président Éblé,

C'est précisément parce qu'il s'inscrit dans le sillon du parcours d'éducation artistique et culturelle suivi par les jeunes, de la maternelle au lycée, que ce passeport a un sens. Il n'est pas une mesure isolée.

La méthode d'élaboration du pass est évidemment déterminante pour sa réussite. À cette fin, nous avons créé une start-up d'État pour le concevoir, de construire l'outil et de déterminer les contours de l'offre dans les prochains mois, en concertation avec les différentes parties prenantes : les futurs usagers d'abord, c'est-à-dire les jeunes, les partenaires potentiels de l'offre, publics et privés, et les collectivités territoriales, bien sûr, nombre d'entre elles ayant déjà lancé des expériences de ce type. Cette méthode de coconstruction est la meilleure voie pour aboutir à un outil en phase avec les usages. Le périmètre de l'offre et le financement seront définis au fur et à mesure de la concertation, en fonction des propositions qui seront mises sur la table par nos partenaires potentiels.

L'objectif est d'aider les bibliothèques à ouvrir « plus ». L'État apportera un accompagnement financier. Un financement supplémentaire est bien sûr prévu, monsieur Hugonet, puisque l'État abondera la dotation globale de décentralisation pour les bibliothèques 8 millions d'euros dès 2018. Je sais que vous vous êtes mobilisée, madame Robert, en faveur de cet objectif, et je vous en remercie. Cependant, tout ne se résume pas à des moyens financiers. L'objectif est également d'aider les bibliothèques à ouvrir « mieux pour devenir ce que j'appelle des « maisons de services publics culturels », c'est-à-dire des lieux qui proposent, comme elles sont déjà nombreuses à le faire, plus que le seul prêt de livres : des services d'aide aux devoirs, des cours de français ou de langues étrangères, des ateliers d'aide à la rédaction de CV. Il s'agit lien étant si important pour la société aujourd'hui. Nous accompagnerons ce mouvement dès l'année prochaine. Les DRAC se rendront disponibles pour réunir les différentes parties prenantes- élus, bibliothécaires, structures sociales et associations locales -et accompagner les projets d'ouverture. : je souhaite que, à la fin de l'année 2018, nous ayons aidé 200 bibliothèques, soit deux par département, à s'engager dans une transformation. Le troisième relais de notre politique culturelle de proximité, c'est le patrimoine, car c'est l'une des ressources culturelles les plus équitablement réparties sur notre territoire. Sur près de 45 000 monuments historiques protégés en France, la moitié se situe dans des communes de moins de 2 000 habitants. Sa mise en valeur peut nous aider à insuffler de la vie là où les commerces ferment, là où les transports en commun se font rares, là où l'exclusion frappe. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur pour avis, j'ai présenté le 17 novembre ma stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, laquelle comprend quinze grandes mesures. Elle s'appuiera sur un budget renforcé. Les moyens dédiés à l'entretien et à la restauration du patrimoine s'établiront à 326 millions d'euros en 2018, soit une hausse de 5 % par rapport à 2017. Un tel niveau n'a jamais été atteint depuis dix ans.

pour la restauration du patrimoine situé dans des communes de moins de 10 000 habitants. Une expérimentation sur la revitalisation des centres-villes anciens est actuellement conduite dans dix-sept villes de France, dans le prolongement des propositions faites par votre ancien collègue, Yves Dauge. Plusieurs ministères participent à cette expérimentation, dont le ministère de la culture, qui y consacrera 9 millions d'euros l'année prochaine. Nous allons conseiller les collectivités concernant leurs plans de restauration patrimoniale, notamment, et le développement de lieux culturels de proximité. Nous allons par ailleurs engager un travail avec les architectes des Bâtiments de France, les ABF, pour faire évoluer leur rôle. Ce point a été soulevé par le rapporteur. Je souhaite qu'ils puissent intervenir davantage en amont des autorisations, qu'ils jouent un rôle de conseil, afin de fluidifier les délivrances. Un groupe de travail réunissant des ABF et des élus sera lancé dans les prochains jours.

Une plateforme est en ligne depuis deux semaines déjà sur le site du ministère de la culture, dans le cadre de la mission qui a été confiée à Stéphane Bern sur le patrimoine en péril. Elle permet aux citoyens de signaler des monuments près de chez eux. Pour conclure sur le patrimoine, qui est un axe prioritaire

créateurs. J'aurais pu commencer par eux, parce qu'il n'y a pas de vie culturelle sans eux et parce qu'ils savent, mieux que personne, établir ce lien de proximité que nous convoitons entre les oeuvres et nos concitoyens. Leur budget sera conforté l'an prochain porté à près de 780 millions d'euros. Il sera marqué notamment par une hausse des crédits en faveur des structures labellisées. Les moyens nouveaux dégagés, à hauteur de 6 millions d'euros, seront réservés aux projets qui touchent les publics et les territoires éloignés : résidences dans des zones rurales ou des quartiers, projets hors les murs, festivals itinérants Pour soutenir la création, nous allons continuer de veiller aux conditions de vie des professionnels. Nous avons trouvé une solution pour compenser la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs. Le Gouvernement a choisi de mettre en oeuvre un dispositif par voie réglementaire permettant aux caisses gérant les prestations sociales des artistes et auteurs de compenser cette hausse.

de prévention de la délinquance, le FIPD, a vocation à en prendre le relais. Nous discutons avec le ministère de l'intérieur la reconduction de son intervention.

portes ouvertes et de visites pour les citoyens dans des lieux dédiés à la création partout en France : établissements publics, mais aussi ateliers d'artiste, galeries, fonds d'art contemporain. Nous allons y travailler.

les musiques et formule dix recommandations. Le ministère organisera dans les semaines qui viennent une concertation rapide avec les organisations professionnelles pour en discuter. J'annoncerai en début d'année les décisions que le Gouvernement aura prises sur cette base. Je souhaite naturellement mettre à profit ce temps de réflexion pour engager une discussion avec le Parlement. Vous le savez, Roch-Olivier Maistre propose la création d'un établissement public, à partir de ce qu'est aujourd'hui le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV. Si une telle mesure devait être adoptée, elle devrait être entérinée dans une loi.

le ministère des affaires étrangères ; vous en avez débattu il y a quelques jours. Nous allons par ailleurs renforcer largement le soutien à la musique française, qui est en pleine effervescence. Nous avons ainsi décidé de doubler l'année prochaine la subvention du ministère au Bureau export. Nous y reviendrons là encore à l'occasion d'un amendement.

Parallèlement à cette initiative, le CNC va réformer son aide aux vidéoclips musicaux, qui sera portée à 3 millions d'euros. C'est une première en Europe, et un soutien important à la filière musicale, à l'heure où 82 % des internautes, des jeunes, déclarent aller sur YouTube pour regarder et écouter des vidéoclips musicaux.

de vous rappeler l'histoire d'un jeune homme, Janek, le narrateur d', de Romain Gary. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il vit des mois terré au fond d'un trou, dans la forêt, parmi les résistants polonais. Dans le cauchemar de la peur, du froid et de l'obscurité, sa survie tient à trois choses : à l'amour de celle qu'il rencontre, à l'amitié de ceux qui l'entourent et à la culture. Il trouve « sa raison d'être », au sens premier, dans les poèmes qu'il lit, dans les airs de piano qu'il part écouter au péril de sa vie et dans la grâce d'un violoniste qui, en quelques notes, fait « sortir le monde du chaos « Au commencement mourut la haine », écrit-il, « aux premiers accords, la faim ».

Vous avez vous-même confié une mission à l'Inspection générale des affaires culturelles, laquelle rendra son rapport à la fin de l'année 2018. il nous semble prématuré d'engager d'ores et déjà des crédits pour choisir un logiciel informatique alors que nous n'avons pas encore réfléchi ensemble aux objectifs.

les moyens du programme « Patrimoines » enregistrent une augmentation de 3,6 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 0,4 %. Comme je l'ai annoncé lors de la présentation de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, j'ai souhaité que les moyens alloués à l'entretien et à la restauration des monuments historiques soient portés à 326 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une hausse de 5 %. Ce niveau sera consolidé chaque année, tout au long du quinquennat. Cela permet notamment la mise en place dès 2018 d'un fonds incitatif et partenarial réservé aux monuments des communes à faibles ressources comptant moins de 10 000 habitants, pour 15 millions d'euros en autorisations d'engagement. À ces moyens s'ajoutent 36 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 26 millions d'euros de crédits de paiement pour le financement des projets d'investissement spécifiques de l'État. En outre, comme vous le savez, la mise en place du loto pourrait rapporter environ 20 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine en péril. Par ailleurs, la mise en place du pass culture est un engagement fort du programme du Président de la République et du Gouvernement. Nous y sommes attachés, car c'est un outil déterminant pour l'accès de la jeunesse à la culture. Il permettra de valoriser l'ensemble de l'offre des établissements culturels de notre pays dans tous les territoires. Il favorisera aussi l'accès

? Je n'ai pas du tout été convaincu par vos propos, madame la ministre. Si j'ai bien compris, le pass culture doit s'inscrire dans le prolongement de ce qu'ont déjà réalisé les départements et les régions. il est absolument essentiel de faire un bilan de ces expériences avant de concevoir le logiciel. À l'école, on m'a toujours appris qu'il fallait d'abord poser un cadre, fixer des objectifs,

Culture ». L'ASTP est alimentée par le produit d'une taxe sur la billetterie, ainsi que par une subvention de l'État et de la Ville de Paris. L'association, gestionnaire de fonds publics perçus pour accomplir ses missions, est donc placée sous la tutelle de ses financeurs et soumise au contrôle économique et financier de l'État. Le modèle de ce fonds de soutien, qui permet un mécanisme de solidarité interne à travers une mutualisation des risques en assurant un taux de garantie aux théâtres privés, est essentiel à la diversité et au dynamisme de création contemporaine du théâtre privé. Or les conditions économiques du secteur du théâtre privé ont connu une évolution qui menace désormais l'équilibre de ce fonds de soutien : stagnation du prix des billets et du financement de l'État, l'ASTP connaît un déficit structurel de 1 million d'euros par an depuis 2010. Après avoir puisé dans sa trésorerie, celle-ci ne lui permet plus aujourd'hui de maintenir sa mission de solidarité dans des conditions raisonnables pour préserver la diversité de création. Alors que ses projections financières ne lui permettent qu'une visibilité à deux saisons, l'ASTP a d'ores et déjà été contrainte de mettre en place des mesures de solidarité plus restrictives. Elle a ainsi fait passer le taux de garantie pour les théâtres privés de 40 % à 35 %. En tant qu'élue de Paris, je vous redis, madame la ministre, qu'il est urgent de renforcer la subvention de l'État pour soutenir le théâtre privé, qui compte 1 000 emplois permanents, sans parler des intermittents. Aujourd'hui, la subvention attribuée au théâtre privé équivaut à 1 % des moyens que l'État consacre au théâtre subventionné- 1 % ! -et à 0,5 % du total des aides de l'État au spectacle vivant, toutes disciplines confondues. C'est vraiment trop peu ! Le présent amendement vise donc à proposer un rattrapage maîtrisé et raisonnable de la subvention de l'État pour préserver durablement ce secteur. J'espère, madame la ministre, monsieur le rapporteur spécial- cher collègue de la Ville de Paris -, que vous saurez le prendre en compte.

des propos ou des éléments attribués au Président de la République, des réformes envisagées. On nous annonce un texte global en 2018, avec, d'après ce que j'ai compris de nos interlocuteurs,

On ajoute ici ou là quelques euros, mais, dans le fond, on a l'impression que le budget pour 2018 est un budget d'attente : avant la réforme avant la réforme d'ampleur attendue, espérée ou crainte, on ne touche pas trop aux équilibres. Pourtant, il va bien falloir y toucher, madame la ministre,

la masse des ressources publiques à répartir entre les sociétés nationales de programme baisse de 1 % par rapport à 2017. Dès lors, on pourrait presque se réjouir de voir progresser légèrement les montants alloués aux opérateurs de l'audiovisuel extérieur. Mais, en réalité, il ne faut pas s'arrêter à la simple arithmétique et il faut observer la situation de ces médias. C'est ce que je vais m'efforcer de faire s'agissant, tout d'abord, de France Médias Monde. Sans doute, la société ne voit-elle pas ses crédits diminuer, mais augmenter de 6,2 millions d'euros, dont 4,4 millions au financement, en année pleine, du programme en espagnol lancé en septembre, conformément aux dispositions du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'État en avril dernier. ce montant, c'est là que le bât blesse, est inférieur de 1,9 million d'euros au montant inscrit pour le financement de ce contrat en 2018. Or l'entreprise ne dispose pas de véritables marges de manoeuvre. Côté ressources, elle est financée à plus de 95 % par des ressources publiques, et les ressources publicitaires, nous l'avions écrit dans nos précédents rapports, sont surestimées. Les prévisions pour 2018, comme celles pour 2017 d'ailleurs, laissent un besoin à financer de l'ordre de 0,6 million à 0,7 million d'euros par an. Nous avions avancé trois pistes pour les rendre plus dynamiques l'alignement dans le cahier des charges des dispositions concernant la publicité de RFI et MCD sur celles de Radio France, l'extension de la diffusion de France 24 et de RFI sur le territoire national, enfin la capacité pour France 24 de rapatrier en interne la régie confiée actuellement à France Télévisions Publicité ou de la confier à une autre structure. J'aimerais savoir, madame la ministre, où nous en sommes sur ces trois dossiers. Côté charges, France Médias Monde a mené une politique drastique de baisse des charges de fonctionnement et a réalisé, il n'y a pas si longtemps, deux plans de départs volontaires pour amincir son pôle radio et financer le lancement de France 24. Elle s'est aussi organisée pour engager un dialogue social sur l'évolution des métiers de journalistes et de technicien, permettant ainsi de vrais gains de productivité. Elle devra absorber cette année les conséquences de l'accord passé par les entreprises de l'audiovisuel et les syndicats sur la prise en compte de l'ancienneté des pigistes, qui n'entrait pas dans les hypothèses du COM. La poursuite des économies devant d'ores et déjà permettre de financer les développements inclus dans le COM, il n'est guère possible d'aller plus loin. La seule solution, sauf à accepter une exécution déficitaire, pourrait être de toucher à la diffusion de France 24 à l'échéance de certains contrats, notamment à New York et Los Angeles, ou de fermer une rédaction régionale de RFI en Afrique. Ce n'est pas acceptable au moment où nos concurrents traditionnels, mais aussi des émergents et des groupes non étatiques- parfois terroristes -engagent des moyens importants au service de stratégies d'influence, dont le principal souci n'est pas toujours la défense des valeurs démocratiques et une éthique de l'information respectueuse de la vérité des faits et de la liberté d'expression des opinions. La seule alternative, et nous partageons en ce sens l'analyse du rapporteur spécial de la commission de finances, consiste à rétablir les crédits de France Médias Monde au niveau inscrit dans le COM. Nous défendrons un amendement de la commission des affaires étrangères en ce sens.

qui prévoit la transformation numérique de l'entreprise, chantier indispensable pour ne pas rester à l'écart de la mutation du marché mondial. Cette évolution est d'autant plus nécessaire que la réalisation des objectifs du précédent plan avait été entravée par une cyberattaque de grande ampleur en 2015. La société doit, par ailleurs, soutenir ses priorités géostratégiques, en première ligne desquelles l'Afrique où la concurrence se renforce et où la diffusion par la TNT devient un objectif majeur. Elle doit également poursuivre sa transition avec la diffusion en haute définition, renforcer sa politique de sous-titrage et la distribution de ses chaînes thématiques. Si les États contributeurs ont souscrit aux objectifs du plan stratégique, ils n'ont pas, pour autant, apporté les ressources nécessaires à son financement, loin de là. Après une légère augmentation de la contribution française en 2017, l'allocation de ressources publiques pour 2018 est inférieure de 1 million d'euros. Cette baisse est une première historique, et cela ne donne pas, hélas, un bon signal à nos partenaires belge, suisse, canadien et québécois, dont la contribution tarde déjà à atteindre le niveau requis. Nous souhaiterions savoir, madame la ministre, si vous avez espoir que ceux-ci puissent réajuster le montant de leur contribution en 2018. Dès lors, la société devra poursuivre son développement, en s'efforçant d'absorber les glissements et indexations contractuelles, en poursuivant ses efforts de réduction des frais généraux, en limitant l'impact sur sa grille de programmes et en faisant prévaloir les priorités du plan stratégique, à savoir l'Afrique et le numérique, à défaut de pouvoir les déployer dans toute leur ampleur. Je conclus, monsieur le président. Au moment où s'engage sur les ondes et dans l'espace numérique une véritable lutte informationnelle, il importe donc que la France soit présente avec ces deux entreprises et qu'elle en assure le développement. Derrière les chiffres, la réalité est tout autre, mais nous avons espoir de vous convaincre et de redresser la situation. Nous souhaitons donc, sous réserve du vote de l'amendement que nous proposons proposons s'agissant de France Médias Monde, et en reconnaissant que ce budget, ainsi corrigé, à défaut d'être celui du plus grand bien pour les opérateurs de l'audiovisuel extérieur sera celui du moindre mal, donner un avis favorable

pour tenir compte de l'évolution des usages et de la nécessité de mieux veiller à l'utilisation de l'argent public. Les efforts demandés à France Télévisions en sont l'incarnation la plus frappante dans ce budget, mais nous nous félicitons, dans ce contexte, qu'ARTE et France Médias Monde voient leurs moyens préservés, de même que l'INA et TV5 Monde. Au chapitre des déceptions, il y a sans doute Radio France : la situation du chantier reste très préoccupante, et nous attendons avec impatience le rapport de M. Weiss pour y voir plus clair. Était-il, dans ces conditions, justifié de préserver Radio France, qui bénéficie d'une hausse sensible de sa dotation de fonctionnement, alors même que les réformes se font attendre ? Notre principal regret tient sans doute à l'absence de préavis qui a accompagné la remise en cause des moyens de l'audiovisuel public. Comme si les impératifs budgétaires avaient primé les considérations culturelles et sur la cohérence d'une politique de l'audiovisuel. Ce regret ne remet pas en cause l'avis favorable que notre commission a donné aux crédits de l'audiovisuel, car il nous semblait essentiel de vous envoyer un message

à l'audiovisuel public, ce qui est loin d'être garanti aujourd'hui. Celle-ci passe par la spécificité de ses contenus et l'indépendance à l'égard des annonceurs. Deuxièmement, les mutualisations doivent être plus radicales que les pistes énoncées par les chaînes : rapprochement des rédactions, fusion des services support, diminution des masses salariales, développement des plateformes numériques communes, remise en cause de certains services ... Seul l'actionnaire a l'autorité de fixer une feuille de route à des entreprises qui ont pris goût à une certaine forme d'autogestion et à une hausse continue de leurs moyens. Troisièmement, cette feuille de route doit être portée par un fort. La nomination d'un patron commun à France Télévisions et à Radio France pourrait constituer une première étape. s'agissant de la révolution numérique, nos sociétés publiques n'ont pas la taille critique ni l'expertise pour mener les investissements nécessaires. Avec le changement de modèle marqué par la délinéarisation, l'État sera bientôt propriétaire de quatre petites sociétés produisant des contenus audiovisuels diffusés d'abord sur internet. Le regroupement doit permettre de financer des contenus d'avenir au lieu d'entretenir des structures du passé. Il y a urgence à changer de modèle. Nous soutiendrons donc ce budget constituant la première étape

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vieillissement du lectorat, fuite des recettes publicitaires, impasse industrielle de la vente au numéro, la presse s'enfonce dans une crise que la vitalité de la presse digitale peine à enrayer. La faute à une rentabilité incertaine, à un partage de la valeur déséquilibré et à la concurrence des nouveaux modes d'information. Sans réaliser de miracle, les aides à la presse représentent un soutien indispensable. Le programme 180 « Presse et médias » de la mission « Médias, livre et industries culturelles » en constitue la traduction budgétaire. En 2018, les aides à la modernisation, à la diffusion et au pluralisme s'élèveront à 119,4 millions d'euros, en légère diminution en raison de la réforme de l'aide au portage. Ces crédits sont complétés par une enveloppe de 131,5 millions d'euros destinée à l'Agence France Presse. Dans un contexte de crise, seul le digital montre une croissance dynamique, mais il ne représente encore en moyenne que 5 % du chiffre d'affaires des éditeurs. L'accélération de la mutation numérique doit donc constituer un objectif prioritaire. Les éditeurs du digital bénéficient d'un soutien des pouvoirs publics qui ne cesse de s'étoffer. Outre le taux super réduit de TVA, les sites d'information politique et générale sont éligibles au Fonds stratégique pour le développement de la presse, qui, avec 27,3 millions d'euros en en 2018, représente le principal soutien à des projets de développement numérique, ainsi qu'au Fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation de la presse, doté de 5 millions d'euros en 2018. Pour autant, les aides indirectes bénéficient encore à 54 % à l'imprimé, et la différence est encore plus nette pour les aides directes : sur 100,2 millions d'euros versés en 2016, 89,5 millions d'euros l'ont été à la presse papier. En réalité, à l'exception des deux fonds précités, l'ensemble des dispositifs de soutien à la modernisation, à la diffusion et au pluralisme sont réservés aux publications imprimées. Vous conviendrez avec moi, madame la ministre, qu'une meilleure répartition entre les publications pourrait être envisagée. L'enjeu est à la fois économique et démocratique : la presse doit avoir les moyens de s'imposer dans l'univers numérique comme la garante d'une information de qualité face à des sites diffusant des contenus pour le moins sujets à caution. J'en viens enfin à la situation de l'Agence France Presse, qui continue d'inspirer les plus grandes inquiétudes. Malgré le lancement d'un plan de relance commerciale ambitieux, son chiffre d'affaires peine à décoller, tandis qu'une politique d'investissement, indispensable mais dispendieuse, a conduit l'Agence à un niveau de dettes de 52,6 millions d'euros à la fin de l'année 2016, auxquels s'ajoute un découvert bancaire de 26,4 millions d'euros. Malgré les efforts réalisés, notamment la signature d'un accord d'entreprise unique, la maîtrise des charges ne peut suffire à dégager les moyens de se désendetter ni d'investir. sans capitaux ni actionnaire, l'Agence ne peut se financer sur les marchés, tandis que le droit européen limite l'intervention de l'État. Malgré ces réserves, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de ce programme.

avis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le programme 334 « Livre et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles consacrera, en 2018, 262 millions d'euros en autorisations d'engagement et 271 millions d'euros en crédits de paiement au livre et aux industries culturelles, soit, à périmètre constant, une augmentation de 2 % en crédits de paiement. C'est au livre et à la promotion de la lecture que profite la quasi-totalité des crédits du programme- 94,4 % précisément -, raison pour laquelle j'y consacrerai l'essentiel de ma courte intervention. Dans ce cadre, 215 millions d'euros correspondent à la subvention pour charge de service public de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information. Je ne m'appesantirai pas sur la description d'une charge budgétaire destinée essentiellement à financer des dépenses contraintes de fonctionnement de ces opérateurs. En revanche, j'aimerais vous interroger, madame la ministre, dans la mesure où la BNF est, aux côtés du Centre national du livre, opérateur du programme de numérisation des livres indisponibles du XX siècle, sur l'avenir du dispositif ReLIRE. Jugé contraire au droit européen par la Cour de justice de l'Union européenne, le 16 novembre dernier, en raison d'une information insuffisante des ayants droit, il n'apparaît pas non plus conforme à la mouture prévue par le projet de révision de la directive du 22 mai 2001, en cours de discussion. Avez-vous bon espoir de faire aboutir la position française sur le sujet ? Dans cette attente, quelle suite est réservée, en 2018, à ReLIRE, dans lequel plusieurs millions d'euros ont déjà été investis ? Dans le temps qu'il me reste, j'évoquerai enfin les 9 millions d'euros de subvention à la HADOPI. Stable, cette enveloppe permettra à l'opérateur de poursuivre sa mission de lutte contre le piratage et de promotion de l'offre légale. Après les déboires budgétaires de l'institution, nous pouvons nous en réjouir. Il n'empêche, la lutte contre le piratage doit s'exercer au plus près des nouvelles pratiques. Que dire dès lors d'un opérateur dont la mission se limite au téléchargement « pair-à-pair », peu en vogue aujourd'hui, sans traiter les ravages du ? La HADOPI elle-même, consciente de ce décalage, a commandé une étude sur les évolutions possibles de la riposte graduée. Les travaux menés en 2015 par Corinne Bouchoux et Loïc Hervé, au nom de notre commission, avaient envisagé un système de sanction plus automatique. Quelles sont les perspectives d'évolution des missions de la HADOPI et, plus généralement, des politiques de lutte contre le piratage dans ce contexte de libéralisation ? Nonobstant plusieurs points de vigilance, que vous trouverez développés dans son avis écrit, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 334 de la mission

Monsieur le président, madame la ministre de la culture, monsieur le président de la commission des finances,

soit une diminution de 13 millions d'euros par rapport aux crédits votés en 2017. Cette baisse des crédits s'explique en réalité par un double mouvement financier : d'une part, le transfert des crédits du ministère de la culture consacrés à l'éducation artistique et culturelle à un programme de la mission « Culture », que nous avons évoqué un peu plus tôt dans la journée, d'autre part, la prise en charge de l'aide à la diffusion du cinéma en région par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. Il convient par ailleurs de rappeler que les crédits de cette mission ne représentent qu'une partie des concours financiers de l'État au secteur des médias, du livre et des industries culturelles. En effet, l'effort financier global s'élèvera à 1,75 milliard d'euros en 2018, grâce au concours des taxes affectées au CNC et au Centre national du livre, le CNL, et aux dépenses fiscales rattachées aux deux programmes de la mission. Si ces chiffres sont rassurants, le secteur est cependant soumis à un double défi : d'abord, la législation et la réglementation ont vieilli et méritent d'être modernisées ; ensuite, la profession est confrontée au défi de la transformation numérique. De vrais engagements ont pourtant été pris au cours des derniers mois pour relever ce défi. D'abord, en septembre dernier, la taxe sur les ventes de vidéos, affectée au financement du CNC, a été étendue aux plateformes de vidéos payantes installées à l'étranger- la fameuse taxe Netflix -et aux plateformes composées majoritairement de vidéos gratuites- la taxe YouTube. C'est une prise en compte lucide de la transformation des pratiques de consommation des médias. Ensuite, dans les mois à venir, le Parlement devra intervenir pour consolider l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, à la suite de la décision d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel.

Soutien aux médias de proximité, Soutien à l'expression radiophonique locale et Compagnie internationale de radio et de télévision. Cette décision n'est pas neutre politiquement. Alors que la liberté de la presse a été plusieurs fois menacée par des attaques terroristes au cours des dernières années, le renforcement des aides financières à la presse est un devoir d'intérêt général. Si les crédits de ce programme sont en diminution de 2,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, à 284,9 millions d'euros pour 2018, ils restent en hausse sensible, à périmètre constant, par rapport aux crédits effectivement consommés en 2016. Les aides à la presse sont donc stables dans le temps, et nous nous en félicitons. Notre groupe y est très sensible, estimant que la défense de nos médias est un secteur stratégique de nos politiques publiques en France et à l'étranger. Sur le programme 334 « Livre et industries culturelles », les efforts de l'État en faveur du développement de la création littéraire et de sa diffusion sont louables : organisation d'un grand débat national sur la lecture, lancement de la deuxième édition de la nuit de la lecture, poursuite des actions prioritaires engagées en faveur du développement du livre, poursuite de la démarche en faveur de l'accessibilité des livres numériques aux personnes en situation de handicap, poursuite de l'adaptation aux enjeux du numérique, Ce budget offre aussi l'opportunité de soutenir plus fermement l'entrepreneuriat culturel, avec l'organisation du forum Entreprendre dans la culture, manifestation parisienne déclinée dans nos régions avec pour but d'aider à la professionnalisation et à la structuration des entreprises culturelles. Je crois que nous pouvons tous saluer cette démarche d'information et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs du secteur. Quant au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », il est marqué par un effort général de réduction des dépenses. C'est un engagement à la rationalisation des moyens de ce secteur, dans la perspective d'une réflexion plus générale sur l'évolution du modèle de financement des médias. Petit bémol cependant, notre groupe remarque que la diminution des crédits de l'audiovisuel pèse principalement sur France Télévisions- 2018 -et que celle-ci n'est pas répartie équitablement entre les sociétés de l'audiovisuel. Cette réduction des moyens a des conséquences lourdes sur la politique audiovisuelle extérieure. La direction de France Médias Monde a ainsi dû revoir sa couverture internationale à la baisse pour réaliser des économies. Cette décision touche à notre diplomatie d'influence française et, de la même manière que notre groupe a salué les efforts de renforcement des moyens du Bureau Export de la musique française et a déposé un amendement à ce sujet, nous attirons votre attention sur l'importance de doter le service public audiovisuel des moyens nécessaires à son action internationale. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission de la culture, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et afin d'encourager les efforts entrepris au cours des derniers mois par le Gouvernement, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera en faveur des crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles », tout en appelant à une certaine vigilance sur notre rayonnement culturel international.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parmi les crédits consacrés à cette mission, je concentrerai l'essentiel de mon propos sur la société France Télévisions, qui bénéficie de plus de 2,5 milliards d'euros pour 2018, soit les deux tiers des moyens alloués au secteur de l'audiovisuel public. Comme on le dit en langage courant, France Télévisions alimente beaucoup la gazette depuis quelques semaines. C'est normal, dira-t-on, qu'un grand média fasse parler de lui, mais, en l'occurrence, ce n'est ni la qualité de tel ou tel programme, ni l'exclusivité de telle ou telle information diffusée sur ses antennes, ni ses succès d'audience qui nous valent autant de remue-ménage autour de cette entreprise. De rapports confidentiels en notes tout aussi confidentielles savamment répandues dans la presse- nous y avons encore eu droit pas plus tard qu'hier -, de critiques pas même voilées à l'endroit de sa tutelle en déclarations fracassantes sur telles coupes telles coupes à venir dans les achats de programmes ou dans les émissions d'information, on ne peut pas dire que la direction actuelle de France Télévisions ménage ses efforts. Sans compter l'intense travail de lobbying déployé auprès de certains de nos collègues ou des syndicats de producteurs ... Non, on ne chôme pas en matière de communication au siège de l'entreprise. Dommage d'ailleurs qu'il n'existe pas d'indicateur de performance en la matière, car il y aurait là précisément matière à satisfaction

à 2,9 milliards d'euros. Mais, bizarrement, ce qui est demandé à l'ensemble de la Nation pour redresser les comptes publics paraît irréalisable pour cette société de service public, plus marquée par la culture de la dépense que par la culture de l'efficacité et de l'innovation. Certes, à la décharge de France Télévisions, il faut reconnaître que l'entreprise évolue dans un univers extrêmement concurrentiel et marqué par des évolutions technologiques profondes. Quelques initiatives ont bien été prises, mais, dans la grande inertie et les errements stratégiques qui caractérisent depuis longtemps cette entreprise, celles-ci n'ont pas toujours été très judicieuses. La création en 2016 de France Info TV, supposée coûter peu d'argent, en est l'illustration. Fruit d'une mutualisation de moyens avec Radio France et, plus accessoirement, avec France Médias Monde, son audience s'avère pâle pour un coût réel qui reste totalement opaque. La comptabilité analytique ne semble pas être le fort de la maison et aucun chiffrage sérieux n'a jusqu'à présent été produit à ce sujet. du secteur, son coût réel serait de 60 à 80 millions d'euros par an, soit plus du double de celui de LCP et Public Sénat réunis, pour une audience inférieure à ces deux chaînes En concurrence directe avec LCI, BFM TV et CNews, on ne s'étonne guère de la faiblesse de son audience, d'autant qu'on peine à voir, en dehors de l'absence de publicité à l'antenne, de grandes différences de contenus avec ces autres chaînes d'information continue. Était-il pertinent de lancer une chaîne linéaire supplémentaire dans un marché déjà saturé ? Difficile de ne pas avoir le sentiment d'une certaine gabegie quand on sait que la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, finance déjà une chaîne d'information de qualité qui s'appelle France 24, mais qui demeure largement inaccessible à celles et ceux qui paient pour qu'elle existe. d'ailleurs fallu batailler ferme en 2013 pour que cette chaîne dispose enfin d'une fenêtre de quelques heures sur un canal de la TNT en Île-de-France. Elle sert désormais aussi de bouche-trou sur le canal de France Info TV entre minuit et six heures du matin quand les programmes de la première s'arrêtent. Bref, France 24, c'est comme une belle chambre, payée plein tarif, mais avec deux lucarnes en guise de fenêtres et sans vue sur la mer ... Trouvez l'erreur Pour en revenir à la gestion de France Télévisions, on peut, comme l'a récemment fait la Cour des comptes, s'interroger sur une présence pléthorique des postes d'encadrement au sein de cette société. Certaines fonctions supports de France Télévisions comme les ressources humaines ou la communication- pour n'en citer que deux -ont des effectifs sans commune mesure avec toute autre entreprise, y compris publique, de moins de 10 000 ETP dans ce pays Cette multiplication insensée de postes d'encadrement impacte terriblement la masse salariale, pour des fonctions qui ne sont pas directement liées à la production et à la diffusion de programmes, le coeur de métier du groupe. Selon le rapport de la Cour des comptes précédemment cité, 191 salariés touchent ainsi plus de 120 000 euros brut par an, et 547 plus de 96 000 euros la grande maison de l'audiovisuel français ne compte pas que des chambres semi-aveugles. Elle comporte aussi, surtout à l'étage France Télévisions, des placards obscurs qui contrastent avec d'autres, bien plus dorés. Dans quelle autre entreprise de communication trouve-t-on un ancien directeur de l'information, démissionnaire depuis le 22 mai dernier, toujours rémunéré par l'entreprise à un niveau de salaire inchangé, pour une mission qui recoupe très largement des fonctions déjà occupées par d'autres cadres de la société ? pourrait paraître presque anecdotique si l'intensification de la concurrence venant d'acteurs mondiaux ainsi que les nouveaux usages et modes de consommation des médias n'appelaient pas au plus vite une réforme en profondeur d'un modèle économique de la télévision publique aujourd'hui à bout de souffle. Même si l'effort budgétaire demandé à France Télévisions ne représente qu'un infime pourcentage de son budget, nous le considérons comme un préalable bienvenu à une réforme d'envergure. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera en faveur des crédits de cette mission. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parce que le monde de la création connaît aujourd'hui une profonde mutation, parce que les créateurs et créatrices doivent être soutenus et leurs oeuvres protégées, parce que l'accès de chaque citoyen à une information fiable et indépendante constitue l'un des piliers de notre démocratie, on ne peut que refuser les grands arbitrages proposés dans ce projet de budget pour la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Nous avons besoin d'évaluer sérieusement les effets de la montée en puissance d'une concurrence internationale féroce pour le monde de la création française. La mise en place de taxes sur le chiffre d'affaires publicitaire des plateformes vidéo pour financer la création audiovisuelle est sans doute une bonne nouvelle. Mais je doute que le seul produit de ces taxes suffise à répondre aux besoins de moyens pour la création française, ni que leur mise en place limite les appétits européens des multinationales qui, avec leurs moyens immenses, sont en train de mettre la main sur tout le marché. Madame la ministre, vous ne prévoyez rien non plus contre la concentration dans la presse et la mainmise de la finance. Aujourd'hui, dix personnes contrôlent 90 % de l'audience des quotidiens, 55 % des télévisions et 40 % des radios. Parmi eux, des vendeurs d'armes, des industriels, des professionnels de la banque et des fraudeurs fiscaux, avec le soutien complice de certains politiques. Il faut maintenant légiférer pour empêcher cette concentration dans les médias et empêcher toute situation de monopole qui hypothéquerait gravement la liberté de l'information. Dans ce contexte, il est inacceptable de proposer une baisse de 2,6 % des aides à la presse, qui permettent justement aux organes de presse encore indépendants de résister et d'exister. Il faut au contraire amplifier ces aides publiques, en les orientant prioritairement vers les titres qui en ont le plus besoin, pour permettre un véritable développement de la presse d'information politique et générale. Dans la lignée du combat que nous menons aux côtés des journalistes et salariés de France Télévisions pour « une télévision publique dont le sens profond est de se libérer des seules règles d'un jeu qui ne serait qu'économiquement profitable et socialement tolérable nous nous opposerons à la saignée budgétaire imposée à France Télévisions par le Gouvernement avec le soutien de la droite sénatoriale. Parce que cela a profondément fragilisé le groupe, nous dénonçons depuis le début la non-compensation des pertes de recettes publicitaires, estimées à 35 millions d'euros,

Vous prévoyez pourtant une baisse sans précédent de la dotation du groupe de 35 millions d'euros, alors que les effectifs n'ont cessé de diminuer, avec un plan de départs volontaires de plus de 500 personnes, puis le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux, soit, dans le contrat d'objectifs 2016-2020, 1 000 suppressions de poste envisagées. De fait, les équipes sont à bout et le service public est en danger. Si les mesures du document de travail du Comité action publique 2022, révélé le 13 novembre, se concrétisaient, le service public audiovisuel serait directement menacé de disparition à court terme.

Sans aggraver la dépense publique, qui semble tant effrayer le Gouvernement, des solutions existent pour trouver de nouveaux moyens pour le service public. Vous pourriez par exemple renforcer la taxe sur les recettes publicitaires des chaînes privées, une manne potentielle à l'heure où celles-ci négocient une troisième coupure publicitaire en soirée Pour cette mission budgétaire, comme pour les autres, la seule ambition du ministère de la culture se résume en un mot : accepter les économies. Pour y parvenir, sous couvert de compétitivité, de recours au privé et de désengagement de l'État, on s'apprête à sacrifier des pans entiers de ce qui fait la force culturelle et de pensée de notre pays. Il est encore temps d'y renoncer : c'est pourquoi nous voterons contre ce budget. La parole

par le secteur public, car c'est lui qui ordonne l'ensemble. On le sait, sans le service public de l'audiovisuel, l'investissement dans la création

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur spécial, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, l'actualité relative aux contours de cette mission me pousse à commencer mon propos en relevant la baisse de 1 % des crédits alloués à l'audiovisuel public. Sur le fond, nous déplorons un repli des moyens affectés à l'audiovisuel public, après une hausse de 100 millions d'euros l'an passé. Sur la forme, nous regrettons le caractère tardif de l'information faite aux bénéficiaires de ce budget- seulement à la fin du mois d'août dernier. Ce manque de visibilité ne permet pas de s'adapter à ces restrictions budgétaires dans de bonnes conditions et viendra contrarier la réalisation des objectifs contractuels. Dans le cas précis du groupe France Télévisions, la baisse s'établit à près de 50 millions d'euros. On regrettera également que cet effort budgétaire ne s'accompagne pas d'un horizon précis. Au-delà de la préservation de ses moyens, France Télévisions a aujourd'hui besoin d'une véritable feuille de route, comme d'ailleurs l'ensemble de l'audiovisuel public français. Je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir de France Télévisions s'inscrit dans le cadre de son identité et de la spécificité de son offre. Il convient de les préserver dans un environnement plus ou moins détaché des exigences de l'audimat à court terme et de la publicité. En effet, la poursuite d'une démarche essentiellement « commerciale », sur le modèle des groupes privés, ne saurait être salutaire et ôterait progressivement, aux yeux de nos concitoyens, la légitimité de son financement public. Nous le savons, le Gouvernement travaille à une remise à plat de l'audiovisuel public. Je rappelle, à cet égard, les réformes structurelles que le Sénat appelle de ses voeux depuis plusieurs années pour ce secteur. Réforme de la gouvernance, du financement, des synergies : autant de chantiers que nous souhaitons pleinement accompagner dans un avenir proche au sein de la Haute Assemblée. Concernant le budget des aides à la presse, force est de constater que ce secteur ne connaît toujours pas le rebond que nous lui souhaitons. La crise se poursuit du fait d'une rentabilité des divers acteurs toujours trop incertaine et d'une concurrence grandissante des nouveaux moyens d'information. Seule la presse digitale parvient à tirer à peu près son épingle du jeu. Elle représente un des uniques leviers de croissance actuels. Mais, là encore, sa rentabilité est fragile du fait des difficultés à capter les recettes publicitaires et de la faiblesse du prix de ses abonnements par rapport aux éditions papier. Notre réflexion doit aujourd'hui se porter sur une meilleure disponibilité, en direction du numérique, des dispositifs existants de soutien à la modernisation. Les aides publiques à la presse demeurent donc plus que jamais indispensables. Celles-ci s'établissent à un niveau à peu près stable pour 2018, autour de 120 millions d'euros. L'Agence France Presse bénéficiera également d'une enveloppe à peu près constante, d'environ 130 millions d'euros. Néanmoins, les difficultés de financement de l'AFP et son avenir suscitent une légitime inquiétude. Le programme 334 « Livre et industries culturelles » présente des crédits destinés, pour l'essentiel, au soutien public au livre et à la lecture. 215 millions d'euros accompagneront la Bibliothèque nationale de France, pour laquelle d'importants investissements sont toujours engagés sur le site Richelieu, et la Bibliothèque publique d'information, rattachée au centre Pompidou. Ces crédits vont également à notre vaste réseau de 16 000 bibliothèques et de points d'accès au livre, l'un des plus étendus d'Europe. En dépit de cette couverture importante- près de 90 % de nos compatriotes -, le nombre d'usagers réguliers de ces structures demeure modeste. Pour l'essentiel, cela s'explique par les horaires d'ouverture de nos bibliothèques, qui présentent un caractère contraignant pour la plupart des personnes. La charge d'une extension de ces horaires repose aujourd'hui essentiellement sur les collectivités territoriales. Un grand nombre d'entre elles se sont déjà engagées dans cette voie. Cet effort a une incidence significative sur la masse salariale. Il convient donc de les accompagner dans cette dynamique visant à permettre à nos concitoyens un accès simplifié à la lecture. Cet enjeu a déjà été mis en exergue par le Sénat et c'était d'ailleurs l'un des engagements de campagne du Président de la République. Vous avez, madame la ministre, confié une mission en ce sens à M. Érik Orsenna. Lors de l'examen des crédits de la mission « Relations

Concernant le marché du livre en France, qui continue de bénéficier d'une protection particulière, son chiffre d'affaires demeure stable. Le secteur se porte plutôt bien et doit pouvoir continuer de se reposer sur un réseau de vente fourni. Le plan Librairie, mis en oeuvre par le précédent exécutif, a fait oeuvre utile, même s'il n'est pas parvenu à enrayer la détérioration continue de ce marché depuis plusieurs années. Il convient donc de sanctuariser les dispositifs de soutien aux libraires, tout comme ceux qui sont destinés aux éditeurs et aux auteurs. À ce titre, la définition d'un nouveau modèle de financement du Centre national du livre devient pressante. En effet, le rendement des taxes affectées au CNL est insuffisant depuis plusieurs années, ce qui conduit à limiter le champ de ses interventions. Enfin, en conclusion de ce rapide panorama, j'évoquerai le cinéma, désormais rattaché à cette mission, et le sursis donné au CNC par le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne pourra percevoir, au-delà du 1 juillet prochain, la taxe sur les éditeurs de services de télévision. Il nous faudra donc d'ici là sécuriser juridiquement ce dispositif générant 300 millions d'euros de recettes. Sur l'ensemble des points soulevés, le groupe du RDSE demeurera vigilant. Il apportera toutefois son soutien aux crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». La parole

public. Notre groupe suivra l'avis des rapporteurs de ces deux commissions. L'effort général de réduction des dépenses demandé aux sociétés de l'audiovisuel public appelle une explication de notre part ; mon propos portera donc sur ce sujet. Il y a un an, la commission de la culture de notre Haute Assemblée refusait d'approuver le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Quelques mois auparavant, le rapport des sénateurs Jean-Pierre Leleux et André Gattolin faisait le constat de la dégradation de la situation financière de l'audiovisuel public, notamment de France Télévisions. Dans ce contexte, il s'avérait indispensable de réduire les dépenses et de rationaliser les moyens. Le précédent gouvernement, en signant le dernier COM de France Télévisions, n'a pas pris en compte les remarques de notre commission. Trois engagements majeurs n'y étaient pas inclus : les effectifs de France 3, la mobilisation de la filière interne de production et la réduction du coût des achats de programmes. Le présent budget est cohérent avec ces réserves. Notre groupe souhaite toutefois préciser qu'il ne peut s'agir que d'une solution d'attente. Une réflexion globale sur la place de l'audiovisuel public dans notre pays doit être engagée. En effet, les usages se sont modifiés avec l'arrivée des géants de l'internet. La diffusion de la création française est mise à mal et l'offre explose. Les supports de lecture se sont diversifiés, le poste de télévision n'étant plus l'écran principal où sont diffusés les contenus. La question du modèle de financement de l'audiovisuel public se pose de façon accrue dans un contexte de dégradation des finances de l'État et alors que les autres ressources sont incertaines, avec, d'une part, le déclin du marché publicitaire et, d'autre part, un retour sur investissement insuffisant en matière de production. Soit, les Français contribuent directement au financement de l'audiovisuel public par l'acquittement d'une redevance, mais ils ont maintenant accès à un large panel de chaînes privées et souhaitent donc que leur participation corresponde à une réelle valeur ajoutée. Certains pays européens se distinguent par la qualité de leur audiovisuel public et la plupart ont déjà engagé des réformes structurelles. La BBC, en Grande-Bretagne, a su maîtriser ses dépenses, en constituant un groupe unique qui regroupe l'ensemble des radios et des télévisions nationales, locales et internationales. Cela lui permet de mutualiser ses moyens et de mobiliser davantage d'investissements. Face aux évolutions technologiques et aux nouveaux usages, c'est le modèle historique de l'audiovisuel public à caractère national évoluant dans un univers peu concurrentiel qui doit être revu. En l'absence de réforme, les médias du service public risquent fort de décrocher. Après un quinquennat de, le Gouvernement semble décidé à faire bouger les lignes, mais pour le moment, madame la ministre, nous n'en sommes qu'au stade des suppositions. Le Parlement, en particulier le Sénat, a un rôle majeur à jouer dans cette réflexion et plusieurs pistes ont été avancées par le rapport d'information de Jean-Pierre Leleux et André Gattolin. L'expérience des dernières années montre qu'il est plus facile de reconduire des crédits que de mener une réforme qui s'annonce d'ampleur. J'approuve donc la demande formulée par notre commission, sur l'initiative de sa présidente Catherine Morin-Desailly, Morin-Desailly, d'un débat qui pourrait être organisé courant janvier 2018 afin d'engager la réflexion et d'éclaircir les intentions du Gouvernement. Mes chers collègues, les défis à relever sont nombreux. Quel modèle économique et financier définir ? Comment réformer la contribution à l'audiovisuel public ? de la publicité- Roger Karoutchi a évoqué quelques pistes de réflexion à ce sujet -et de la prise en compte de l'audimat ? Enfin, peut-on conserver un modèle de gouvernance, dont l'indépendance est contestable ? En 2018, notre groupe participera activement à cette réflexion, afin que notre audiovisuel puisse relever les défis de demain et remplir la mission éducative, culturelle et citoyenne qui lui revient. La parole est à M.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget pour 2018 de la mission « Médias, livre et industries culturelles » est un budget de transition

Notons que les aides à la presse, qui représentent 120 millions d'euros en crédits de paiement en 2018, sont marquées, cette année, par une diminution des aides à la diffusion et un maintien du niveau des aides à la modernisation numérique. La santé de la presse est notamment mesurable à ses ventes, qui sont en décroissance constante : depuis 2011, la baisse des ventes des quotidiens nationaux atteint un peu moins de 10 %, alors que les ventes numériques augmentent de plus de 42 % sur la même période.,

qui subit une baisse de plus de 5 %. Le journal le plus impacté semble être, dont la diffusion chute de 17 %. Au-delà des chiffres,

Ce besoin de réformes concerne également l'audiovisuel public. Le législateur devra intervenir avant le 1 juillet 2018 pour consolider l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, à la suite de la décision d'inconstitutionnalité rendue le Conseil constitutionnel le 27 octobre dernier. Les économies demandées sont au coeur de l'actualité et je voudrais attirer votre attention sur un point symptomatique des difficultés de notre pays à se réformer. De 2012 à 2017, le gouvernement de l'époque a proposé l'augmentation du budget alloué à France Télévisions. Cette évolution n'aura pas permis d'engager de véritables réformes structurelles ni de repenser son mode de fonctionnement dans son ensemble. Aujourd'hui, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2018, l'audiovisuel public doit réaliser, contraint et forcé, des économies à hauteur de 47 millions d'euros qui, hier encore, paraissaient inconcevables. Preuve par l'exemple que, oui, un budget en baisse n'est pas forcément un mauvais budget s'il s'appuie sur des réformes structurelles à la hauteur des enjeux. Certainement, nous pouvons regretter que ces réformes n'aient pas été menées plus tôt et qu'une fois encore, le précédent gouvernement ait eu recours à la facilité d'une augmentation des crédits budgétaires sans engager les réformes structurelles. Il est désormais indispensable de les faire.

ou non sur la redevance. Concernant la question de la redevance et, de manière plus large, celle du financement de l'audiovisuel public, nous ne pouvons que souhaiter que le Gouvernement s'inspire fortement des recommandations de l'excellent rapport de nos collègues Leleux et Gattolin de 2015, qui présentait des pistes sérieuses et crédibles pour pérenniser les financements, sans peser sur les finances publiques. C'est le cas notamment du système de financement dit « à l'allemande », pour lequel le groupe Union Centriste a indiqué, à de nombreuses reprises, son intérêt, en particulier au regard du critère de justice fiscale : ce système permet en effet de faire participer l'ensemble des foyers au financement de l'audiovisuel public. Pour conclure, les crédits du programme « Livre et industries culturelles » sont stables. Mention honorable en ce qui concerne le financement de la Bibliothèque nationale de France, qui participe au redressement des comptes publics, puisque sa dotation 2018 diminue modérément de 2,5 %, et le maintien

Ne perdons jamais de vue l'enjeu principal de toute réforme : l'adaptation à l'évolution des habitudes de consommation de nos concitoyens en lien avec les nouvelles technologies.

Les réformes sont sûrement un mal nécessaire, mais à trop forte dose, ne risque-t-on pas de tuer le malade ? » Soyons justes, cette inquiétude est légitime, mais elle n'est souvent que l'alibi du conservatisme ! En attendant ces réformes, que nous appelons de nos voeux, le groupe

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'information est la bataille du XXIe siècle. Avec l'avènement et la profusion du numérique, elle est, encore plus qu'auparavant, un enjeu central de puissance et d'influence. Instrument décisif, elle peut même influer le cours des événements de manière inattendue et irréversible, comme de nombreux faits récents l'attestent. C'est pourquoi le rôle des médias classiques, singulièrement de la presse écrite, est encore plus essentiel aujourd'hui et est une responsabilité collective, qui appelle de notre part vigilance et exigence. vigilance et exigence. Lutter contre les tendances à la « post-vérité », rétablir les faits à travers des articles pédagogiques, mais aussi apporter au lecteur une mise en perspective de ces faits sont des missions fondamentales. Pour ce faire, la presse a besoin de moyens. En premier lieu, la situation financière de l'AFP, malgré les réformes d'ampleur déjà engagées, demeure préoccupante. Elle affronte une concurrence mondiale exacerbée, mais le marché de la vidéo, en pleine expansion, peut représenter une piste de réflexion intéressante.

les aides au pluralisme et à la modernisation constituent pourtant une priorité ; il est d'ailleurs dommage que le fonds stratégique pour le développement de la presse subisse une légère baisse. En effet, la presse a besoin d'un appui affirmé et, surtout, d'une véritable réforme structurelle visant à assurer son modèle économique, à protéger ses éditeurs, à garantir le pluralisme et à conforter l'indépendance des journalistes et des rédactions. Il serait donc intéressant que le Gouvernement formule une véritable stratégie de soutien à la presse, afin de définir clairement les axes sur lesquels il compte insister à l'avenir. À l'échelle européenne, la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse dans le cadre de la directive visant à réformer le droit d'auteur est à soutenir, eu égard aux nouveaux usages numériques. Je tiens à saluer la position ferme de l'exécutif sur ce sujet, en espérant vraiment qu'elle convainque l'ensemble de nos partenaires. En ce qui concerne le volet « Livre et industries culturelles », il est marqué par une transformation profonde de périmètre, surtout pour le livre et la lecture publique, du fait de transferts de crédits au programme 224.

À cet égard, le contexte actuel semble favorable pour renforcer la politique de lecture publique, et spécialement le rôle des bibliothèques, pour lesquelles vous connaissez mon attachement. Je me réjouis donc de l'annonce du Gouvernement, qui vise à augmenter de 8 millions d'euros la

et du jazz, le CNV. Mes chers collègues, on le voit, pour garantir le pluralisme et la diversité, les outils de régulation sont désormais vitaux. Certains existent et doivent être confortés, mais je suis certaine que de nouveaux restent à inventer. Très

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j'ai pu vous présenter, un peu plus tôt, les grands axes de ma politique culturelle, que je veux d'émancipation, pour ceux qui se sentent aujourd'hui sur le bord de la route, et de cohésion, à l'heure où il arrive à notre société de douter. Les médias, les livres et les industries culturelles y jouent évidemment un rôle crucial, parce qu'ils sont, d'ores et déjà, ancrés dans le quotidien de la plupart de nos concitoyens. À l'heure du numérique À l'heure du numérique et alors que quelques grands acteurs dominent le marché, notre principale responsabilité est de veiller à la diversité des oeuvres et des contenus, auxquels nos concitoyens ont effectivement accès, et à l'indépendance de ceux qui les diffusent.

Je ne reviendrai pas sur les pistes de travail qui ont été rendues publiques le mois dernier, alors qu'elles n'avaient pas vocation à l'être. Je le répète devant vous : le document qui a été publié n'était pas une ébauche de feuille stratégique, mais un document de recensement des principales propositions mises sur la table ces dernières années. Ces pistes de travail seront enrichies par de nouvelles discussions et par les propositions que j'ai demandé aux sociétés de l'audiovisuel public de me faire. Nous assumons notre volonté de transformation. Nous avons engagé un travail de recensement et de réflexion, mais je prendrai le temps de la concertation. J'ai reçu, un à un, la majorité des dirigeants la semaine dernière et je recevrai les autres cette semaine. La volonté de transformation est largement partagée, partagée, parce que l'avenir du service public en dépend. Nous sommes donc dans un dialogue on ne peut plus constructif. Les enjeux sont multiples. Il s'agit d'abord d'adapter notre modèle de régulation aux nouvelles réalités du secteur. La législation et la réglementation ont vieilli. Elles ont été conçues dans les années quatre-vingt, à une époque où il n'y avait que six chaînes de télévision, diffusées par voie analogique. Trente ans après, tout a changé : le nombre de chaînes, la profusion des contenus, le numérique, l'arrivée des géants de l'internet, les écrans connectés, partout et tout le temps. Notre législation a été modifiée à de nombreuses reprises, mais elle reste marquée dans son inspiration par ce temps qui fut celui de la rareté, auquel a succédé l'ère de l'abondance, dans laquelle nous sommes dorénavant.

Au niveau national, nous avons lancé une consultation sur l'évolution de la réglementation en matière de publicité à la télévision. Les services du ministère sont en train d'examiner les réponses. Nous avons aussi ouvert le chantier de la réforme de la chronologie des médias, qui est une priorité pour adapter notre modèle aux nouveaux usages et sécuriser l'avenir de notre système de financement des oeuvres. J'ai confié une mission de médiation à M. Dominique D'Hinnin pour faire aboutir les discussions au sein de la profession, qui étaient bloquées depuis trop longtemps. Je lui ai donné un maximum de six mois pour trouver un nouvel accord. À défaut, le Gouvernement prendra ses responsabilités et n'exclut pas de proposer une solution législative, en lien étroit avec le Parlement qui a déjà travaillé sur cette question. Des avancées importantes ont eu lieu sur la contribution des acteurs numériques au financement de la création, comme l'a rappelé Mme Mélot. Je pense notamment à l'entrée en vigueur, au mois de septembre, des taxes dites YouTube et Netflix, qui élargissent la taxe vidéo affectée au CNC à toutes les plateformes. J'ai enfin annoncé, il y a quelques semaines, que le Gouvernement s'engageait franchement en matière de lutte contre le piratage. Comme l'a indiqué Mme Laborde, le piratage des oeuvres et des contenus est un fléau que nous devons combattre par tous les moyens. J'y travaille avec mon collègue Mounir Majhoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, ainsi qu'avec l'ensemble des ministères concernés. Le programme de travail est clair : nous devons évaluer l'existant,

comme l'a indiqué Mme Robert, en faveur de la protection du droit d'auteur et de la reconnaissance du droit voisin au profit des organismes de presse- c'est l'une des clés pour assurer un modèle économique viable à la presse en ligne. j'ai participé aux négociations sur la directive Services de médias audiovisuels, dite SMA, qui est actuellement en discussion entre les institutions européennes. Nous espérons que ces négociations aboutiront au premier semestre 2018. La transposition de cette directive devrait avoir lieu prochainement en France : elle ouvrira la possibilité d'une refonte de la régulation audiovisuelle, qui est issue de la loi de 1986. En parallèle de ces chantiers de modernisation légale et réglementaire, nous allons engager une réforme de fond de l'audiovisuel public. Elle repose sur une vision, l'affirmation de missions prioritaires et une méthode de transformation. Une vision, d'abord. Les médias de service public jouent un rôle indispensable dans le paysage médiatique et dans notre société en général. Je le redis devant vous avec force. À l'heure où les sources de contenus se multiplient et où l'information circule de façon abondante, ils ont une valeur de référence pour nos concitoyens. Ils offrent un repère essentiel. Nous voulons conforter leur rôle, dans un environnement qui évolue fortement.

informer, cultiver, divertir », l'audiovisuel public est aujourd'hui un acteur de premier plan en matière de soutien à la création et à la diffusion de la culture, d'information, de services de proximité et de rayonnement international de la France. Dans le contexte des profondes mutations que nous connaissons, l'audiovisuel public a sa carte à jouer pour affirmer sa singularité par rapport non seulement aux chaînes privées, mais aussi aux nouveaux géants du numérique. Premièrement, il doit faire le pari de la création et proposer des programmes qui se distinguent dans un univers d'offre surabondante. Deuxièmement, il doit être à la pointe de l'offre numérique et multicanal pour s'adapter aux nouveaux usages et se tourner davantage vers les jeunes générations. Troisièmement, enfin, il doit développer une stratégie ambitieuse à l'international. Ce positionnement stratégique nécessite de profondes transformations, dont certaines sont déjà engagées par les équipes dirigeantes, comme l'a rappelé M. Assouline. Le Gouvernement est déterminé à accompagner ces changements. Je voudrais aussi dire un mot de la méthode. Ces défis devront, vous le savez, être relevés dans un contexte contraint pour les finances publiques, le Gouvernement s'étant engagé, en toute responsabilité, dans une politique de redressement des comptes publics. L'audiovisuel public doit contribuer à l'effort collectif, ce qui suppose d'ajuster les dotations prévues dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus par le précédent gouvernement. Le budget de l'audiovisuel public sera de 3,9 milliards d'euros l'année prochaine. L'effort d'économies demandé est réel, je ne le conteste pas : il s'élève à 36 millions par rapport à 2017 et 80 millions par rapport aux

Le budget 2018 reste supérieur à ceux de 2016 et de 2015. Monsieur Ouzoulias, en ce qui concerne les magazines d'information de France 2, je note que la présidente de France Télévisions a d'ores et déjà annoncé que leur fréquence serait maintenue. j'ai fixé quatre impératifs stratégiques à court terme : soutien à la création et à l'offre culturelle ; information de référence ; transformation numérique de l'offre pour accélérer les mutations et s'adresser davantage aux jeunes ; rayonnement international de la France.

représente un effort important que je tiens à souligner. Je reviendrai sur la question de France Médias Monde à l'occasion de la discussion des amendements. Pour préparer l'avenir, je souhaite que l'audiovisuel public

le financement ; la gouvernance. En ce qui concerne la réflexion sur le périmètre des missions et l'efficacité de leur mise en oeuvre, elle fait actuellement l'objet d'un travail interministériel, associant mon ministère à ceux de l'économie et des comptes publics, j'ai demandé aux sociétés de l'audiovisuel public de me faire des propositions, qu'elles m'ont rendues à la mi-novembre. Cette réflexion se poursuivra jusqu'au début de l'année 2018. À ce stade, le travail porte notamment sur les coopérations et les synergies, ainsi que sur les meilleures complémentarités qui peuvent être trouvées entre les acteurs du secteur, à l'image de ce qui a été engagé avec France Info. Monsieur Gattolin, l'information est au coeur des missions de service public de France Télévisions et de Radio France : il est donc logique qu'un canal d'information en continu fasse partie de leur offre. Certains parmi vous considèrent qu'il faut regrouper tout ou partie des différentes sociétés de l'audiovisuel public. Si nous n'écartons aucune piste pour l'avenir, je vous indique qu'à ce stade, rien n'est arrêté. Ce débat peut avoir lieu et ce sera le cas le moment venu. la transformation du secteur devra s'accompagner d'un débat sur son financement. Pour ce qui est de la contribution à l'audiovisuel public, sujet que vous avez mentionné, monsieur Lafon, aucun impératif financier ne justifiait une réforme à très court terme. La priorité de ce projet de loi de finances pour 2018, vous le savez, est la réforme de la taxe d'habitation. Néanmoins, à moyen terme, l'évolution des usages pose la question du rendement de cette contribution et de l'équité entre contribuables. Ainsi, comme le ministre de l'action et des comptes publics et moi-même l'avons déjà dit, je souhaite qu'un débat soit ouvert autour, notamment, d'un élargissement de l'assiette.

Le dernier chantier de transformation concerne la gouvernance de l'audiovisuel public. C'est un corollaire indispensable aux autres réformes et nous connaissons les limites du système actuel. Je souhaite que l'on ouvre le sujet, comme le Président de la République s'y est engagé pendant la campagne et comme le Premier ministre me l'a demandé dans sa lettre de mission. Cela concerne, d'une part, les contrats d'objectifs et de moyens, dont les dates ne sont pas alignées, ce qui complique l'exercice par l'État de son rôle d'actionnaire commun, et, d'autre part, les modes de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public. Sur ces deux dossiers, comme sur tous ceux que je viens d'évoquer, je serai évidemment à l'écoute de vos propositions. Je tenais à prendre un peu de temps pour vous présenter ces sujets, car vous l'aurez compris, ce sont des chantiers décisifs, qui traduisent l'ambition forte que nous portons pour les médias de service public et qui doivent préparer leur avenir. Je voudrais, à présent, vous exposer les principales orientations de notre budget pour la mission « Médias, livre et industries culturelles ». À périmètre constant par rapport à 2017, les moyens de cette mission seront quasiment stables l'année prochaine. S'agissant du soutien de la presse- vous l'avez rappelé, monsieur Laugier, madame Jouve -, le budget pour 2018 sanctuarise nos deux priorités, monsieur Ouzoulias, qui sont le coeur du soutien public à la presse. En effet, les aides au pluralisme sont intégralement maintenues et tous les dispositifs d'aide à l'innovation et à la transformation numérique sont préservés. Pour ce qui est de la filière de la distribution de la presse, nous devons naturellement tenir compte des évolutions rapides de ce secteur. Ainsi, les moyens de l'aide au portage diminuent en 2018, en cohérence avec l'évolution des volumes. Les aides à la distribution sont maintenues. Et pour préparer l'avenir de la filière, nous avons confié une mission de réflexion à Gérard Rameix, ancien président de l'Autorité des marchés financiers.

au contrat d'objectifs et de moyens. Nous avons, par ailleurs, engagé une réflexion prospective avec l'AFP sur ses projets, ses investissements technologiques et le développement de sa marque à l'international. Nous souhaitons accompagner le développement des projets de l'AFP, qui est l'une des trois principales agences de presse au monde et qui est, en effet, madame Robert, Le budget pour 2018 réaffirme par ailleurs notre soutien aux radios locales. Les moyens du fonds de soutien à l'expression radiophonique sont confortés à 31 millions d'euros, un niveau historique. J'en viens aux industries culturelles. Pour ce qui est de la musique, j'ai eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure le rapport de Roch-Olivier Maistre et le soutien à l'export. Je voudrais simplement rappeler que nous avons maintenu les deux crédits d'impôt pour la musique et pérennisé l'aide à l'innovation. Pour ce qui est du livre,

l'intention de Mme Robert. L'une de nos grandes responsabilités est de veiller à la bonne application de la loi sur le prix unique du livre, ce que je suis engagée à faire sur tous les canaux, physique et numérique. Quant au dispositif « ReLIRE », que vous avez évoqué, madame Laborde, la France soutient sa sécurisation au niveau européen, dans le cadre de la directive Droit d'auteur. Je me suis déplacée à Bruxelles, la semaine dernière, et je vois, cette semaine, le vice-président de la Commission européenne, M. Andrus Ansip. le sujet lors de notre conversation. Je profite, enfin, de l'occasion qui m'est donnée ici pour vous dire que je partage les interrogations suscitées par l'amendement voté ici même, il y a quelques jours, à propos du label LiR, destiné aux librairies indépendantes. En effet, faute d'une concertation préalable, ses conséquences n'ont pas été, à mon sens, entièrement mesurées. S'il était maintenu en l'état, cet amendement pourrait avoir, entre autres, pour effet de décourager certaines collectivités à maintenir l'exonération fiscale qu'elles accordent aux librairies indépendantes. Il me semble donc préférable d'en rester aux critères actuels, dans l'attente d'une évaluation du label LiR, créé il y a dix ans maintenant, évaluation qui pourrait être conduite dans les prochains mois.

pour atteindre 3 millions d'euros. Les crédits d'impôt pour le cinéma, l'audiovisuel et les jeux vidéo sont, par ailleurs, intégralement préservés, après la forte revalorisation des deux dernières années. Ils ont permis de réaliser deux objectifs majeurs pour notre économie : la relocalisation des tournages et des studios en France l'augmentation du volume de production dans deux secteurs clés pour l'exportation, les séries et les dessins animés. Dans le seul secteur de l'animation, l'emploi a crû de 15 % en une seule année. C'est dire que dans l'ensemble des domaines, la création française est soutenue de façon pérenne. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, voilà l'essentiel des orientations de notre budget pour l'audiovisuel public et pour la mission « Médias, livre et industries culturelles » pour l'an prochain. Vous l'aurez compris, dans chacun des secteurs, notre budget est à la fois garant des principes fondamentaux du modèle culturel français et vecteur de la transformation dans laquelle nous voulons engager notre pays. Nous allons procéder

Nous proposons de porter la hausse à 1 million d'euros pour doter cet organisme des moyens nécessaires. Le Bureau Export de la musique française accompagne chaque année près de 300 artistes français à l'international et assure leur présence sur plus de 80 projets professionnels. Cette mesure vise donc à assurer le rayonnement international de la culture française. Elle répond aussi à la transformation de l'industrie musicale, sous l'effet des nouvelles technologies numériques.

qui est d'éviter de dépouiller les uns pour essayer de combler la pénurie des autres ! Là, en l'occurrence, la victime, c'est France Télévisions, qui a déjà payé beaucoup. Je vous rappelle que ses crédits ont baissé de 0,4 % et ses effectifs de 6,2 %, baisse à laquelle s'ajoute une perte importante de recettes publicitaires due aux réformes de 2009 et de 2016.

est devenue extrêmement difficile. Je le dis après Roger Karoutchi, une société a fait énormément d'efforts et nous avons l'impression que c'est toujours l'opérateur le plus vertueux qui est le plus pénalisé ! Or nous avons vraiment besoin de ce rayonnement français à l'international, pour des tas de raisons, notamment économiques. Une chaîne publique en français, qui n'est malheureusement pas encore assez diffusée, est indispensable, surtout au regard des efforts que font nos concurrents partout dans le monde, y compris sur des terres où nous avions, jusqu'à présent, un quasi-monopole, comme l'Afrique. Beaucoup d'autres compagnies et sociétés étrangères s'impliquent. Nous sommes dans un contexte extrêmement concurrentiel et nous avons donc besoin de rendre les moyens à France Médias Monde. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à

? Je comprends les préoccupations qui ont motivé ces amendements. Dans le contexte actuel, l'audiovisuel extérieur joue un rôle essentiel pour apporter dans le monde un point de vue français sur l'actualité. Pour continuer à remplir cette mission, notre audiovisuel extérieur fait face à des défis considérables, vous l'avez noté, marqués par l'intensification de la concurrence dans le paysage des médias internationaux, la révolution numérique et l'évolution des modes de diffusion. En parallèle, France Médias Monde doit assurer le financement en année pleine de France 24

la plus forte de tout l'audiovisuel public. Je souhaite apporter quelques précisions sur ce budget abordé par M. Karoutchi et par Mme Garriaud-Maylam. France Médias Monde a d'ores et déjà travaillé à l'élaboration de son budget pour 2018 en tenant compte de la réduction de 1,9 million d'euros de ses crédits par rapport au montant prévu au contrat d'objectifs et de moyens. Le projet préparé dans ce cadre, communiqué aux administrations et qui sera débattu en conseil d'administration à la fin du mois de décembre, ne remet pas en cause sa capacité à assurer son rayonnement mondial, ne préempte aucun choix stratégique pour l'avenir et ne fragilise pas sa soutenabilité financière. En revanche, France Télévisions et Radio France assument des missions tout aussi essentielles, comme l'information, la promotion de la culture et le soutien à la création. Elles doivent elles aussi investir dans le numérique. De ce fait, il n'est souhaitable ni de revoir encore à la baisse les crédits de France Télévisions, à laquelle des efforts sont d'ores et déjà demandés, demandés, ni d'ajuster la dotation de Radio France, sauf à fragiliser l'activité de l'entreprise et à remettre en cause le retour à l'équilibre de ses comptes en 2018. En définitive, le projet de loi de finances pour 2018 proposé par le Gouvernement résulte d'un équilibre entre les contraintes et les priorités des différentes sociétés dans un contexte où il leur est demandé à toutes de participer à l'effort collectif de redressement des comptes publics. Je ne souhaite pas que cet équilibre soit modifié. Pour l'ensemble de ces raisons,

emplois sont le produit de la diffusion audiovisuelle. Or le principal investisseur, c'est France Télévisions. Et vous voulez affaiblir tout cela ! Moi, ! Je pense qu'il faut réaffirmer ici que nous soutenons tout l'audiovisuel public. Nous ne choisissons pas là où on va prendre pour donner ailleurs au moment où vous parlez-

absolument nécessaire d'accompagner la décision de réabonder le budget à hauteur de 1,9 million d'euros. C'est vrai- M. Assouline a raison -qu'il est toujours regrettable de déshabiller l'un pour habiller l'autre.

rassemblent plus de 100 millions d'auditeurs et de téléspectateurs mesurés dans moins du tiers de leur pays de diffusion. Les trois médias du groupe cumulent 35 millions de visites dans leur environnement numérique chaque mois- c'est une moyenne pour 2017 -, dont près de 40 % sur les offres en langue étrangère. Il est ainsi utile que la France puisse poursuivre son rayonnement dans le monde à travers les médias indépendants, notamment pour des personnes aujourd'hui connectées leur téléphone portable ou leur tablette. C'est aussi grâce à ces médias que les Français établis hors de France gardent un lien avec notre pays,

et Mme Garriaud-Maylam ont un objectif extrêmement louable. Au sein de notre commission, nous avons été très nombreux à souligner l'excellent travail de l'audiovisuel extérieur et les problèmes auxquels il se trouve

le Gouvernement. À ce stade de l'année, il faut mesurer que France Télévisions va faire un effort de plus de 47 millions d'euros d'économies- sans doute même 75 millions d'euros si l'on tient compte des hausses des coûts exogènes, contrats

à partir du budget pour 2018 entre l'audiovisuel public traditionnel : Radio France, France Télévisions, FMM et ARTE - on n'a pas beaucoup parlé d'ARTE, qui fait un excellent travail. Cette meilleure répartition et cette grande attention, madame Garriaud-Maylam, à notre audiovisuel extérieur ne peuvent passer

et dire un certain nombre de choses. Je regrette, madame la ministre : si vous m'aviez dit que vous aviez sur vous le chéquier gouvernemental pour trouver 2 millions d'euros de plus, on ne les prendrait à personne ! Nous sommes à budget contraint. Sauf que FMM travaille son budget en

l'enjeu, pour les années qui viennent, est de définir une nouvelle trajectoire qui soit « ambitieuse », c'est-à-dire qui nous remette sur la voie du respect de nos engagements internationaux, mais aussi aussi « crédible », ce qui suppose de consacrer des ressources plus importantes à cette politique. C'est à l'aune de ces éléments que nous avons examiné les crédits 2018 de l'aide publique au développement. La définition d'une nouvelle trajectoire est en effet indispensable, tant la France est éloignée du respect de ses engagements internationaux. L'objectif,

et l'aide britannique, le double. Cette divergence des trajectoires française, allemande et britannique est frappante, mais elle est aussi préoccupante, monsieur le ministre. Le montant des dons octroyés par la France est particulièrement inquiétant. Nous pouvons donc nous réjouir que le Président de la République ait récemment pris l'engagement, devant l'Assemblée générale des Nations unies, d'atteindre un objectif intermédiaire de 0,55 % d'APD d'ici à la fin du quinquennat. Plus précisément, cette augmentation de l'aide devrait notamment porter sur l'aide bilatérale, qui est un meilleur outil d'influence et dont la part a diminué au cours des dernières années. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 traduit en partie cette ambition, avec une augmentation importante des crédits de la mission

Cette trajectoire appelle cependant notre vigilance. Tout d'abord, l'exécution doit être en phase avec les crédits votés. Cet indicateur est révélateur du degré d'ambition accordé à cette politique, qui a tôt fait d'être considérée comme une variable d'ajustement de l'exécution budgétaire.

Nous estimons que les impératifs budgétaires de l'été 2017 pouvaient justifier cette mesure d'économie par rapport au budget du précédent gouvernement, mais les choix présentés au Parlement sont désormais ceux de l'actuelle majorité gouvernementale. Les crédits de cette mission doivent être sanctuarisés. À ce titre, les efforts réalisés pour améliorer la sincérité du budget vont dans le bon sens. Par ailleurs, nous notons que l'effort budgétaire est centré sur la fin du budget triennal. Ce choix est un facteur de risque pour la mise en oeuvre concrète de la programmation. Nous serons vigilants sur son respect. Enfin, pour atteindre l'objectif fixé pour 2022, il faudra aller plus loin et maintenir une trajectoire ascendante sur l'ensemble du quinquennat, voire accentuer cet effort. Il pourra être nécessaire d'écrire cette nouvelle trajectoire dans une loi de programmation de l'aide publique au développement, qui fixe l'effort financier de l'État jusqu'en 2022 et réaffirme nos priorités.

rapporteur spécial de la commission de finances, Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, après le premier de cordée, Yvon Collin, je vais, pour ma part, vous présenter les crédits pour 2018 et les points qui ont particulièrement retenu notre attention. les ressources que consacre la France à l'aide publique au développement en 2018 sont en augmentation. Les crédits de la mission connaissent, en effet, une hausse de 100 millions d'euros environ, laquelle est toutefois entièrement absorbée par l'augmentation de la contribution de la France au Fonds européen de développement. Les autorisations d'engagement diminuent de 30 %, mais cette baisse ne fait que refléter la traditionnelle irrégularité de leur montant au sein du programme 110, en fonction du rythme de reconstitution des différents fonds multilatéraux. Le produit des taxes affectées- taxe sur les billets d'avion et taxe sur les transactions financières -est quant à lui gelé à 800 millions d'euros environ. Enfin, les crédits du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », qui, comme son nom l'indique, retrace uniquement des prêts, sont en hausse de 760 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 260 millions d'euros en crédits de paiement, si l'on exclut les opérations exceptionnelles de l'an dernier.

de développement, l'AFD, qui, vous le savez, est l'opérateur pivot de notre aide bilatérale et qui est engagée sur une trajectoire d'augmentation de 4 milliards d'euros de ses engagements et de 400 millions d'euros de ses dons entre 2015 et 2020. Les crédits budgétaires de l'agence augmentent par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Plus précisément, les crédits permettant à l'AFD d'accorder des dons sont en hausse de 67 millions d'euros en autorisations d'engagement, pour atteindre 400 millions d'euros environ. Par ailleurs, les crédits permettant de « bonifier » les prêts, c'est-à-dire d'abaisser directement le taux d'intérêt proposé aux bénéficiaires de ses concours, connaissent une augmentation de 55 millions d'euros. En outre, l'AFD bénéficie de la « ressource à condition spéciale », prêt de long terme de l'État à un taux extrêmement bas qui lui sert également à accorder des prêts concessionnels. Les crédits correspondant aux activités courantes de l'AFD sont stables. En définitive, le niveau des autorisations d'engagement est en ligne avec la trajectoire de croissance de 4 milliards d'euros de ses

le Parlement a décidé, l'an dernier, d'affecter 270 millions d'euros à l'AFD à partir des recettes de la taxe sur les transactions financières. L'article 19 du présent projet de loi de finances revenait sur cette affectation et attribuait cette somme au Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, qui finance essentiellement de l'aide multilatérale.

Nous soulignons, au passage, que la débudgétisation des dépenses du FSD, qui représentent un quart des crédits d'aide publique au développement, est problématique. Ce procédé nuit au contrôle du Parlement et s'apparente à une variable d'ajustement pour les gestionnaires de la mission.

Le futur contrat d'objectifs et de moyens de l'agence, défini pour la période 2017-2020, sera l'occasion de la préciser et de définir les moyens qui l'accompagneront.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les principaux éléments budgétaires, qui ont déjà été présentés. Notre commission a pris acte de la légère progression des crédits prévue pour 2018

Cet engagement nous permettrait enfin de réduire un peu l'écart avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, deux pays qui ont bien pris conscience des enjeux essentiels qui s'attachent à cette politique. Je veux d'abord faire une remarque relative à l'organisation de notre expertise internationale. La rationalisation La rationalisation de cette organisation a débuté en 2014, sur l'initiative du Sénat, mais n'est pas achevée. La Cour des comptes a plaidé, cet été, dans un référé, pour un rapprochement entre Expertise France et un opérateur qui n'avait pas été fusionné en 2014, Civipol, actif en matière de sécurité intérieure, de protection civile et de gouvernance. En effet, les deux organismes se font actuellement parfois concurrence ou sont conduits à présenter des offres conjointes, qui supposent des montages parfois trop complexes. Selon nous, le rapprochement des deux entités devra se faire en respectant l'esprit de la réforme de 2014, une volonté de simplification et de plus grande efficacité, afin de promouvoir l'expertise française dans le secteur devenu très concurrentiel, mais essentiel, que constitue la coopération technique internationale. d'autres opérateurs pourraient et devraient également être concernés par un rapprochement avec Expertise France, pour permettre à l'offre française d'être encore plus forte. Reste à réfléchir aux modalités concrètes de cette nouvelle étape de la réforme initiée en 2014. Je remercie notre président d'avoir proposé à la commission travail sur cette question importante. Pour faire bref, il s'agit de mieux expertiser, de mieux évaluer, pour aider plus. Ma seconde remarque portera sur l'une des dimensions de l'approche globale dans les pays en crise, celle de l'action humanitaire, qui rencontre un vrai succès. Je sais que c'est l'une de vos priorités, monsieur le ministre. Ainsi, le fonds d'urgence humanitaire, principal instrument du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay en matière d'action humanitaire et de stabilisation, sera abondé, en 2018, autour de 30 millions d'euros, ce qui constitue une nette progression par rapport à 2017. Toutefois, dans ce domaine aussi, nous restons très loin des budgets de nos partenaires européens. On entend parler d'un objectif de 100 millions d'euros, qui serait d'ailleurs raisonnable. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser que la hausse prévue des crédits d'APD dans les années à venir bénéficiera également à cette dimension essentielle de notre action ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le ministre, mes chers collègues, le Président de la République a annoncé une remontée de l'aide au développement à 0,55 % du RNB au terme du quinquennat. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit également une croissance de 16 % des crédits de la mission « Aide publique Les moyens de l'Agence française de développement, l'AFD, seront également en hausse dès 2018. Toutefois, cette hausse ne compense pas l'annulation de crédits budgétaires effectuée en juillet dernier, représentant une coupe de 136 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 118 millions d'euros en crédits de paiement. Dans ce contexte, je veux faire deux remarques. D'abord, pour atteindre l'objectif fixé, il aurait sans doute fallu prévoir davantage d'autorisations d'engagement dès 2018. La mise en oeuvre de projets bilatéraux financés par des dons, type d'interventions que nous souhaitons voir se développer, demande en effet plusieurs années. À défaut de cet apport de crédits dès 2018, il est indispensable que l'AFD mette à profit ce délai pour se renforcer dans des secteurs dont la coopération française s'est relativement désinvestie du fait de la modestie des crédits en dons disponibles depuis de nombreuses années. Je pense à l'éducation, aux services sociaux, mais aussi, par exemple, à l'agriculture ou encore à la maîtrise de la démographie. Dans ces domaines, l'« équipe France » du développement ne fait plus forcément référence face à ses partenaires européens et aux puissances émergentes, même dans les pays d'Afrique francophone. Les équipes de l'agence devront ainsi accomplir, en 2018, un travail en profondeur pour préparer la progression des financements. Cette augmentation devra intervenir dès l'année prochaine, sans quoi il semble peu probable que la trajectoire financière annoncée par le Président de la République puisse être tenue. En effet, il faut une augmentation totale d'environ 1 milliard d'euros d'APD supplémentaire chaque année pour atteindre le niveau annoncé, que nous n'avons plus connu depuis 1995. Les crédits affectés à l'AFD devront également pouvoir bénéficier en partie à Expertise France, par le biais de relations plus étroites entre les deux opérateurs, de manière à renforcer la coordination et l'efficacité globale de notre « équipe France » du développement. Ma seconde remarque portera sur le rapprochement entre l'AFD et la qui s'est traduit par la mise en place toute récente d'un véhicule d'investissement commun, doté de 600 millions d'euros, pour développer les projets d'infrastructures. Il s'agit notamment- vaste programme ! -de tenter de rattraper notre retard sur la Chine, qui a réalisé de nombreuses infrastructures lourdes en Afrique au cours des dernières années. Si nous ne pouvons qu'approuver cette orientation, qui contribuera à rendre la France plus visible dans cette région du monde, il faut toutefois souligner que la priorité reste bien de créer les conditions du développement par des projets d'une taille adaptée au contexte local dans les zones les plus déshéritées. En d'autres termes, il est sans doute très utile de construire un pont ou un échangeur routier dans telle capitale de l'Afrique de l'Ouest, mais si, pendant ce temps, les habitants du nord du Mali ou des alentours du lac Tchad ne disposent pas de services capables d'entretenir une voirie minimale, ils continueront à rester à l'écart du développement, et ces régions resteront des foyers d'instabilité pour leurs pays et pour le monde. Vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre.

je vous remercie, Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans notre monde en crise, il n'y a pas de sécurité sans développement. C'est dire l'importance vitale des crédits que nous examinons.

Nous vivons sur le souvenir des années 80, quand notre aide publique au développement était de 0,6 % du revenu disponible brut, ce qui nous permettait d'agir tous azimuts.

À l'inverse, l'Allemagne fait le choix clair d'un financement massif d'une expertise internationale très bénéfique à ses entreprises, tandis que le Royaume-Uni sait se concentrer sur des territoires géographiques bien plus circonscrits, notamment en Afrique orientale, allant jusqu'à mettre fin à son aide à l'Inde lorsqu'il n'y trouve plus son intérêt. Et, pour soutenir leurs priorités, ces deux pays versent trois fois plus de dons que nous.

400 millions de jeunes de 15 à 24 ans en 2050. Il est impératif que ces jeunes puissent recevoir une éducation de base et, pour un nombre suffisant d'entre eux, un enseignement supérieur de qualité. Il est également nécessaire que l'économie crée assez d'emplois pour absorber ce flux important. À défaut, ce sera l'instabilité, avec un chômage massif, des migrations toujours plus importantes et, probablement, un renforcement des extrémismes. Que faut-il en déduire pour notre aide au développement ? D'abord, il est impératif de remettre l'éducation au centre. Comment justifier que la France se soit désengagée de l'éducation en Afrique francophone ? Comment avons-nous pu laisser l'école publique y perdre tant de terrain ? l'Agence française de développement augmente progressivement son aide bilatérale à l'éducation, mais les montants des subventions restent trop faibles. Sur le plan multilatéral, entre 2014 et 2018, l'engagement de la France pour le Partenariat mondial pour l'éducation, qui a fait la preuve de son efficacité, s'est élevé à 36 millions d'euros, pendant que le Royaume-Uni participait à hauteur de 335 millions d'euros.

le multilatéral, malgré sa complexité, a son utilité, mais encore faudrait-il que nos financements soient en ligne avec nos objectifs et nos intérêts actuels. Ainsi, monsieur le ministre, comment comptez-vous redonner à l'éducation l'importance qui lui revient au sein de notre politique d'aide au développement ? Par ailleurs, si les tendances actuelles se poursuivent, les économies subsahariennes ne devraient créer que la moitié des emplois nécessaires pour permettre à ces 400 millions de jeunes de trouver un emploi d'ici à 2050. Nous devons donc tout mettre en oeuvre pour contribuer à créer un tissu véritablement dynamique et dense. À cet égard, je souhaite saluer l'annonce faite par le Président de la République à Ouagadougou la semaine dernière de la création d'un fonds africain pour les petites et moyennes entreprises. Il est impératif que cet outil ait pour priorité le soutien à des entreprises innovantes, mais aussi intensives en main-d'oeuvre. Il serait également souhaitable qu'il puisse servir de levier à une meilleure coopération des entreprises africaines avec nos PME, lesquelles peuvent notamment faire valoir leur expertise en matière de croissance verte. Ainsi, monsieur le ministre, au moment où le Président de la République vient d'annoncer une redéfinition de notre politique d'aide au développement,

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la semaine dernière, à l'occasion de son déplacement à Ouagadougou, le Président de la République a réaffirmé son « engagement d'avoir une France au rendez-vous du défi du développement ». Pour être à ce rendez-vous, la France va devoir déployer de nombreux efforts, comme cela a déjà été souligné par plusieurs des orateurs précédents. La France aime se donner en exemple

soit 6 milliards d'euros supplémentaires. Cet objectif est ambitieux, mais nous devrions pouvoir l'atteindre.

Président de la République a déclaré vouloir franchir une « nouvelle étape » consistant, pour la France, à se mettre « en situation d'agréger l'aide multilatérale, l'aide d'autres puissances européennes, pour être plus efficace » et « poursuivre les projets dont les Africains ont besoin ». Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous en dire un peu plus sur les contours de cette proposition innovante ? Par ailleurs, le chef de l'État a indiqué vouloir renforcer l'évaluation de l'APD afin que cette dernière réponde davantage aux besoins du terrain. Il faut aussi se féliciter de la concentration de notre APD sur l'Afrique et sur les pays les moins avancés. À cet égard, des propositions intéressantes ont été formulées par le Président de la République, qu'il s'agisse du soutien prioritaire aux programmes visant à la scolarisation des

Je me réjouis que l'Assemblée nationale ait adopté un amendement visant à rétablir l'affectation d'une fraction de la taxe sur les transactions financières- les fameux 270 millions d'euros. Il s'agit d'une excellente initiative que nous soutiendrons. Une partie de l'aide bilatérale française demeure liée. Elle est gérée par la direction générale du Trésor, la Réserve pays émergents- prêts très concessionnels -, et par le Fonds d'étude et d'aide au secteur privé- au secteur privé- dons, études de faisabilité, etc. La mise en oeuvre de ces financements est assurée par Natixis, qui agit au nom et pour le compte de l'État.

ou CICID, le 30 novembre 2016, le précédent gouvernement avait chargé l'AFD de compléter « sa gamme de produits destinés au secteur privé dans les pays bénéficiaires de l'aide française, notamment pour contribuer à la réorientation des investissements privés vers l'économie résiliente et à basse émission de gaz à effet de serre ». Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser les effets de cette réorientation ?

sont ? Dans leur avis budgétaire, mes collègues Jean-Pierre Vial et Marie-Françoise Perol-Dumont suggèrent un « rapprochement opérationnel plus poussé » entre l'AFD et Expertise France afin que ce dernier « apparaisse davantage comme un partenaire naturel pour les projets initiés par I'AFD

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quel bel objectif que l'aide au développement, qui désigne l'ensemble des ressources fournies aux pays pauvres dans le but de favoriser leur développement économique et d'améliorer le niveau de vie de leurs habitants en luttant contre la pauvreté. Il s'agit d'un objectif que nous défendons tous ici. En 1970, les pays de l'OCDE se sont engagés à porter leur effort d'aide au développement à 0,7 % de leur produit national brut. cinquante ans après, peu d'États ont réussi à respecter leur engagement. Notre pays atteint difficilement les 0,38

Cette promesse se traduit-elle dans ce projet de loi de finances ? La réponse est non. Si une augmentation de 100 millions d'euros est bien inscrite, elle dissimule l'annulation, cet été, de 136 millions d'euros de crédits. Ainsi, cette hausse s'apparenterait plutôt à une perte de 36 millions d'euros. Dès lors, pourquoi se priver d'une rentrée fiscale d'environ 3 milliards d'euros en abandonnant l'intégration des transactions faites en une journée dans l'assiette de la taxe sur les transactions financières ? La réponse se situe certainement dans l'opération de séduction menée actuellement auprès des établissements boursiers de Londres. Cela peut s'avérer utile, mais au détriment de nos engagements internationaux qui apparaissent alors moins attrayants

courant jusqu'en 2020, il faudrait s'attendre à une brusque augmentation de l'ordre de 1,5, puis 2,4 milliards d'euros, en 2021 et en 2022. On peut très bien y croire. Cependant, avec une croissance annuelle estimée à 1,7 % par an, une part de 0,55 % du RNB en 2022 représente 14,8 milliards d'euros.

Il est vrai que seul un tiers des sommes consacrées à l'aide publique au développement est inscrit en loi de finances. Toutefois, ce sont bien ces crédits qui impulsent une marque forte.

De plus, il est urgent de revoir la forme de notre aide au développement, qui se concentre de plus en plus sur les prêts et les aides liées, plutôt que sur les dons. Ainsi, la dette des pays pauvres est un gros problème tant pour les États bénéficiaires que pour les États développés. En effet, le recours au prêt grève à long terme les capacités d'investissement et de développement locales

laissant ces pays très vulnérables au moindre choc. Nous en connaissons de nombreux exemples. Certes, les pays développés comme le nôtre accordent des réductions de dettes, mais ils diminuent concomitamment le montant du reste de leur aide au développement.

du fait d'un manque d'alimentation, de soins et d'eau. Autant de tragédies que l'aide au développement devrait concourir à empêcher. En cohérence, le groupe CRCE ne votera pas ce budget

d'abord à l'affirmation de plus en plus forte d'une jeunesse nombreuse, dynamique et informée, qui ne peut plus se satisfaire ni de la gouvernance parfois défaillante des États- qui ne date pas d'hier -ni d'une aide au développement élaborée souvent de manière unilatérale par les bailleurs. C'est bien à cette jeunesse exigeante que le Président de la République s'est efforcé de s'adresser lors de son déplacement en Afrique, la semaine dernière. Pour contribuer à répondre aux aspirations légitimes de cette jeunesse, il me semble impératif de réinvestir- plusieurs l'ont dit avant moi - le champ de l'éducation, y compris celui de l'enseignement supérieur, afin d'éviter que ces jeunes ne doivent systématiquement quitter leur pays pour se former correctement.

Deuxième évolution à prendre en compte, la montée des désordres écologiques, au premier rang desquels le réchauffement climatique. Il en découle, pour les pays en développement, un impératif au moment où ils mettent en place leurs infrastructures économiques, ils doivent prendre d'emblée le chemin d'une croissance soutenable. Cette priorité a été, me semble-t-il, parfaitement intégrée par l'AFD, par Expertise France, et par un certain nombre d'entreprises françaises également en mesure d'y contribuer.

Car nous n'avons pas toujours su, autant qu'eux, définir précisément nos intérêts et articuler en conséquence nos priorités. Très bien ! Actuellement, deux impératifs me semblent s'imposer à nous le premier est de tout mettre en oeuvre pour stabiliser le Sahel afin de pouvoir y réduire à terme une présence militaire très coûteuse ; le second, qui est transversal, est de mieux faire jouer les synergies entre la coopération, la promotion de nos entreprises et le développement de notre commerce extérieur.

et de réponse aux crises », dotée de 100 millions d'euros par an, dont le Sahel constitue l'une des quatre régions de mise en oeuvre. Cet instrument, très attendu, que notre commission avait appelé de ses voeux, a suscité un véritable engouement de la part des ONG. Il s'est toutefois avéré que les procédures de l'Agence française de développement ne permettaient pas de mettre en place des projets de développement dans un délai aussi rapide que souhaité. Il nous reste donc du chemin à parcourir pour articuler avec efficacité l'action humanitaire, la stabilisation et les projets de développement dans les pays en sortie de crise.

l'aide publique au développement est un impératif de justice et de solidarité internationale, mais c'est aussi une composante de notre politique d'influence. Néanmoins, force est de constater, comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, que nous avons échoué depuis quarante ans à remplir nos engagements internationaux en la matière : l'aide publique française n'a jamais dépassé 0,6 % du revenu national brut, contre un objectif fixé à 0,7 % par l'assemblée générale de l'ONU en 1970.

Face à ces défis, nous saluons l'initiative du Gouvernement, conformément aux orientations données par le Président de la République, de remettre la France sur la voie du respect de nos engagements. intermédiaire de 0,55 % du RNB en 2022 nous semble réaliste et l'augmentation de 7 % des crédits la mission « Aide publique au développement » est un bon signal dans ce sens. Notre groupe regarde favorablement cette évolution, mais restera vigilant quant au respect effectif de cet engagement. Dans un contexte budgétaire contraint, la tentation est souvent de considérer l'aide au développement comme une variable d'ajustement. D'autres pays, comme la Chine, en ont au contraire en ont au contraire fait une composante essentielle de leur diplomatie d'influence, en Afrique notamment, avec un volontarisme politique fort et un effort financier conséquent, appuyé sur de puissants opérateurs. Nous pensons également qu'il faut changer de logique dans notre approche de l'aide au développement. Elle constitue certes un impératif de solidarité, mais elle est aussi et surtout un investissement. Un investissement dans l'avenir, un investissement dans la réussite, chez elle, d'une jeunesse qui s'abîme trop souvent dans une course folle vers nos rivages. Un investissement pour que la prospérité, demain, ne soit plus dans ces pays un rêve d'ailleurs, mais une réalité concrète. Avec cet objectif à l'esprit, il faut penser notre aide au développement d'une façon plus large, à la fois dans la définition des bailleurs, dans les types de projets financés et dans le pilotage des fonds. En ce qui concerne les bailleurs, nous devons améliorer l'articulation entre l'État, les collectivités locales, les ONG et les entreprises ou fondations privées, en fonction des expertises de chacun. par exemple, l'accord signé en octobre 2016 entre la fondation Bill et Melinda Gates et le groupe AFD pour financer des projets communs en Afrique subsaharienne dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'innovation financière et la sensibilisation au développement. Ce type d'accord permet des effets de levier importants et allège la tension sur les budgets nationaux. S'agissant des objectifs de l'aide au développement, nous voyons d'un bon oeil la convergence des processus « objectifs du développement durable » et « financement du développement » au cours des dernières années, sous l'égide des Nations unies. Ce rapprochement entre aide au développement et développement durable s'est matérialisé lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, à Addis-Abeba, en juillet 2015. Le programme d'action d'Addis-Abeba, adopté à son issue, a envoyé un message fort sur l'importance du climat et de son intégration dans l'ensemble des politiques de développement. Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations sont des menaces importantes qui touchent l'ensemble des composantes- économique, sociale et politique Les projets visant à atténuer leurs effets devront être mieux soutenus. Nous saluons la création d'une « facilité d'atténuation des vulnérabilités et de réponse aux crises » par le groupe AFD en 2017. Enfin, sur le pilotage des fonds, deux divisions nous apparaissent structurantes et gagneraient à être éclaircies. Je pense tout d'abord à la division entre aide bilatérale et aide multilatérale. Elles n'ont pas la même signification politique ni la même efficacité. ensuite à la division des crédits entre deux programmes budgétaires distincts, pilotés par deux ministères différents. Cet émiettement conduit à multiplier les instances de coordination et fait perdre à notre politique d'aide au développement à la fois lisibilité et efficacité. Sous réserve de ces points de vigilance, et en espérant, monsieur le ministre, que vous pourrez tenir compte de nos pistes de réflexion, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera ces crédits, qui amorcent une remontée en puissance bienvenue de notre aide au développement.

près de 815 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées. Chaque jour, 16 000 enfants meurent avant d'avoir pu vivre, faute d'accès aux soins. Malgré la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement, requalifiés en objectifs de développement durable, beaucoup reste à faire. La perspective démographique de 9 milliards d'hommes d'hommes d'ici à 2050, conjuguée à celle d'un changement climatique certain, invite la communauté internationale à se mobiliser encore davantage en faveur de la lutte contre la pauvreté. Nous ne pouvons le nier, le développement constitue aussi un enjeu géopolitique fort. La crise migratoire touchant l'Europe depuis plusieurs années rappelle cette réalité. L'afflux de réfugiés inquiète un grand nombre de citoyens européens, dont certains pensent à tort qu'embrasser l'idéologie des extrêmes aux élections nationales et locales ouvrirait la voie à des solutions. Le président Macron l'a rappelé mardi dernier, au Burkina Faso, l'Europe a peur d'être « submergée de migrants au risque de la xénophobie ». Cette crise offre un avant-goût de ce que pourrait être notre lendemain, au sein de l'Union européenne : une vague de réfugiés climatiques issus de pays concernés par le réchauffement qui n'ont pas les moyens ni le niveau de développement suffisant pour retenir leurs populations. Déjà, en 1981, à Paris, à l'occasion d'une conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, le président François Mitterrand disait

ans plus tard, plus que jamais aujourd'hui, c'est une évidence : ce qui se passe là-bas nous impacte ici. Aussi les pays les plus riches doivent-ils porter des politiques de développement ambitieuses. Au niveau mondial, l'effort est indéniable. En effet, avec un montant de 142 milliards de dollars en 2016, l'apport global des pays du comité d'aide au développement de l'OCDE a connu son plus haut niveau historique. Mais qu'en est-il de la France ? Nos collègues rapporteurs de la mission ont donné tous les chiffres, mais permettez-moi, néanmoins, d'en rappeler quelques-uns. La France, cinquième contributeur, tient ses engagements. Mais avec 0,4 % pour 2017, le fameux objectif d'une aide au développement fixé à 0,7 % du revenu national brut n'est pas atteint. Nous pourrions le regretter si le projet de loi pour 2018 ne replaçait pas les crédits dédiés au développement sur une trajectoire ascendante. C'est une bonne chose. le chef de l'État a d'ailleurs confirmé l'ambition de porter le montant de l'aide au développement à 0,55 % du RNB en 2022, lors de son récent déplacement en Afrique. C'est un message fort. Nous le savons, la majeure partie des crédits de cette mission est consacrée justement à l'Afrique.

tous les défis- démographiques, économiques, sociaux, culturels. Nous devons y porter toute l'attention qu'exige notre avenir commun. J'observe toutefois que l'effort apporté aux pays les moins avancés n'est pas encore conforme aux objectifs pourtant réaffirmés par le plan d'action d'Addis-Abeba de 2015 et par l'Agenda 2030. Comme vous le savez, monsieur le ministre, remplacer les dons par les prêts, c'est faire peu de cas de la capacité de ces pays à lever des ressources domestiques ou à attirer des investisseurs étrangers. Ne le nions pas, les pays les moins avancés sont dépendants de l'aide publique. Et l'Agence française de développement devrait veiller à un meilleur fléchage de ses projets. j'ajouterai que la France contribue également au développement par son action extérieure. À cet égard, le sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu la semaine dernière à Abidjan envoie un signal fort, avec l'ambition affichée par le président de la Commission européenne de mettre en oeuvre un plan d'investissement de plus de 44 milliards d'euros destiné à l'Afrique d'ici à 2020. Reste à en connaître les modalités. Monsieur le ministre, malgré les réserves que je viens de formuler, parce que les crédits consacrés à l'APD sont orientés à la hausse et parce que l'aide publique au développement n'est qu'une part du soutien que la France et ses partenaires apportent aux pays les plus fragiles,

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, par les temps qui courent, voir une augmentation de 11 % sur un programme budgétaire n'est pas monnaie courante ! C'est bien pourtant ce que représente la hausse de 100 millions d'euros budgétisée pour le programme 209. Sommes-nous en train de nous positionner sur une trajectoire nous permettant d'atteindre le jalon international de 0,7 % du revenu national brut consacré à la solidarité internationale ? Pas du tout, hélas ! Un décryptage des chiffres s'impose, pour ne pas persister dans l'insincérité budgétaire. Alors qu'Emmanuel Macron présente son premier projet de loi de finances, rappelons-nous le précédent quinquennat François Hollande avait fait de l'augmentation de l'aide publique au développement une promesse de campagne. C'est pourtant durant son quinquennat que l'aide de la France a le plus baissé, tombant même en dessous de la moyenne des pays du comité d'aide au développement de l'OCDE. L'APD représente aujourd'hui 0,38 % de notre revenu national brut, alors qu'elle « pesait » encore 0,50 % en 2010. Laisserons-nous l'histoire se répéter ? Emmanuel Macron Emmanuel Macron s'est engagé, y compris devant l'Assemblée générale des Nations unies, à porter l'APD à 0,55 % du revenu national brut d'ici à 2022- objectif est déjà loin d'être ambitieux, alors que six de nos partenaires européens ont, eux, atteint l'objectif onusien de 0,7 %. Or le premier budget qu'il présente ne place pas clairement la France sur une trajectoire permettant d'atteindre cet objectif. milliards d'euros supplémentaires seraient nécessaires d'ici la fin du quinquennat ; ce n'est donc pas de 100 millions d'euros par an qu'il faudrait augmenter ce budget, mais de plus d'un milliard. On est donc très loin du compte De surcroît, cette hausse de 100 millions d'euros qui nous est annoncée est trompeuse, car elle intervient alors que le budget de l'aide au développement a été coupé de 136 millions d'euros durant l'été La hausse des crédits pour 2018 est ainsi inférieure au montant annulé en 2017 ... Le projet de budget triennal 2018-2020 est trop modeste pour rétablir la trajectoire ; il serait

sur cinq ans, une montée en puissance qui pourrait permettre à la France de tenir ses engagements. La taxe sur les transactions financières est un levier important. Dans le contexte du Brexit, je comprends qu'il faille ménager l'attractivité de la place de Paris. Mais augmenter le taux de taxation de la TTF de 0,3 à 0,5 % ne ferait que placer la France à égalité avec le Royaume-Uni Par ailleurs, augmenter la fraction des recettes de cette taxe allouées à l'APD ne nuirait en rien à la finance française, et aurait un impact significatif sur le financement du développement.

Elle n'a même cessé de baisser de 2010 à 2016, jusqu'au rebond du budget pour 2017, rebond réel, salué comme tel, mais rebond tardif et insuffisant. Il n'est donc pas question, ici, pour moi, de faire la leçon au Gouvernement. Pour autant, comment ne pas pointer le décalage entre les discours du Président de la République, aux Nations unies en septembre, en Afrique la semaine dernière, et la réalité du budget que vous nous présentez ? Décalage il y a, en effet, puisque le président Macron avant moi, l'ont beaucoup dit -que d'ici la fin de son quinquennat, l'APD française serait portée à 0,55 % du revenu national brut. Or- cela a été dit par plusieurs des orateurs qui m'ont précédé -le budget pour 2018 n'inscrit pas la France dans cette trajectoire. Pour atteindre les 0,55 %, il faudrait en effet faire passer notre aide de 8,6 milliards d'euros à près de 15 milliards d'euros, soit 1,2 milliard d'euros de plus par an pendant cinq ans. C'est dire si nous en sommes loin, comme nous sommes aussi très loin, et depuis trop longtemps, des fameux 0,7 %, ce chiffre qui fait consensus au niveau international et que d'autres pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark ou la Norvège, Au-delà du budget lui-même, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite ajouter quelques éléments structurels sur notre politique d'aide au développement, qui n'ont pas à voir avec vos décisions- vous êtes en place depuis six mois seulement -, mais qui correspondent à des travers qu'il faut continuer à essayer de corriger dans les années qui viennent.

Les pays les plus pauvres, eux, ne bénéficient que d'un quart de l'aide française, les autres destinataires étant notamment des pays émergents comme la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. La faiblesse de la part des dons dans l'APD française oriente non seulement cette aide vers les pays les plus solvables, mais elle obère nos capacités d'intervention dans les situations de crise ou de post-crise, malgré le travail remarquable accompli par le centre de crise et de soutien. Il est donc plus nécessaire que jamais, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, de continuer à essayer de rééquilibrer notre aide en faveur des dons. Deuxième élément structurel sur lequel je souhaiterais attirer votre attention : la question de l'aide bilatérale et de l'aide multilatérale. Je connais l'inclination des parlementaires français en faveur de la première.

d'un véritable pilotage coordonné et centralisé des aides multilatérales, certaines étant gérées par Bercy, d'autres par le Quai d'Orsay. Le Royaume-Uni, lui,

sur l'aide humanitaire. Elle reste dramatiquement trop faible en France : 2 % de notre APD lui sont consacrés, soit environ 60 millions d'euros en 2017, alors que l'Allemagne lui consacre 4,4 % de son APD, et le Royaume-Uni plus de 10 %.

la plus grande déception est due à votre décision de revenir sur la mesure votée l'an dernier par le Parlement, consistant à taxer les opérations intrajournalières, les fameuses transactions, à partir du 1 janvier 2018 : vous renoncez ainsi à des recettes qui auraient pu atteindre jusqu'à 4 milliards d'euros par an. Au-delà de cet aspect financier, qui n'est pas négligeable, vous renoncez ainsi à une mesure symboliquement très forte, puisqu'elle consiste à taxer la spéculation financière pour financer la solidarité internationale. Un mot, pour conclure, sur les associations, les fameuses ONG, autrement dit la société civile : elles sont des acteurs irremplaçables de l'aide au développement. Elles prennent des risques, elles sont réactives, elles innovent, elles agissent là elles agissent là où d'autres ont du mal à intervenir. L'aide française aux ONG n'est pas suffisante. Le président de la République précédent avait pris l'engagement d'augmenter beaucoup l'aide publique au développement transitant par les ONG ; je ne doute pas que vous aurez à coeur de tenir cet engagement. La part de l'APD française qui transite par les ONG est de 3 % environ ; la moyenne des pays de l'OCDE est de 16 %. 16 %. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, depuis 2012, des efforts ont été engagés ; ils sont insuffisants, je le répète. J'espère vraiment que le gouvernement auquel vous appartenez continuera dans cette voie. Pour l'heure, le budget que vous nous présentez ne nous semble pas

certains orateurs l'ont dit, et je partage complètement leur analyse - : l'aide publique au développement est un instrument de solidarité, mais aussi un instrument d'influence, et un instrument de gestion globale des crises.

acteurs du développement sur la scène internationale est remis en question, en raison d'une baisse continue de nos moyens, qui se

consistant à porter l'aide publique au développement de 0,38 à 0,55 % du PIB d'ici à 2022. Cet engagement a été pris devant l'Assemblée générale des Nations unies, pas n'importe où,

nous préparer à cet horizon. C'est ce que nous commençons à faire, certes modestement, mais la courbe est inversée avec le budget que je vous présente pour 2018 au nom du Gouvernement. Pour arriver à ce montant et à ce niveau, il faut définir une trajectoire. Je suis assez sensible à l'idée, développée tout à l'heure par le rapporteur spécial Yvon Collin, de créer quelque chose qui pourrait ressembler à une loi de programmation

que les dispositifs mis en oeuvre pour accorder cette priorité sont relativement pervers : pour pouvoir assurer cette priorité d'ordre géographique envers les 17 pays les plus pauvres, il faudrait faire davantage de dons que de prêts.

propose une augmentation des fonds de 20 % dans le domaine humanitaire. C'est une amorce, mais une amorce significative, l'objectif étant que nous soyons au rendez-vous des différents événements. Par exemple, le fonds de stabilisation

en utilisant la « facilité vulnérabilité » issue du Fonds de solidarité pour le développement. Cette " facilité vulnérabilité " est un outil tout à fait efficace pour engager ce type de politiques. dernier thème- je réponds ainsi aux préoccupations du président Cambon - : notre action pour l'éducation et pour la santé, c'est-à-dire pour les deux vecteurs où la qualité française et la spécificité de nos interventions sont généralement au

une bonne articulation entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale, singulièrement lorsqu'il s'agit d'aide multilatérale dans le domaine communautaire. Cette dernière constitue un instrument puissant pour nous aider à

qui nous permettra d'être au rendez-vous des engagements pris par le Président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai pu constater que ces orientations avaient le soutien quasi unanime de votre assemblée ; je vous en remercie.